La séance est reprise. La parole est à madame Hamel Gacquerre pour une mise au point, au sujet d'un vote. Allez-y, chers collègues. Oui tout à fait, il s'agira en fait de modifier les votes. Donc je vous dis nominativement les changements de vote. Il en a. 5h. Oui, il faut le dire, faut le dire. Très bien, je vais le faire de suite, je vous remercie. Alors il s'agit en effet de l'explication de enfin de la CMP pardon concernant le projet de loi. ENR donc le scrutin numéro 125. pour. 5. Rectification, pour le sénateur font qui votera contre. Pour Catherine Morin-, Desailly qui s'abstiendra Sonia de la Provoté qui s'abstiendra. Le sénateur qui s'abstiendra et le sénateur Maurey qui s'abstiendra.

Oui, merci monsieur le président, il s'agit d'une mise au point sur le scrutin public nu numéro 120. Mon collègue Philippe Bas souhaitaient voter pour. Acte est donné de votre mise au point ce sera publié au Journal officiel et figurera dans l'analyste politique des scrutins concernés. L'ordre du jour appelle le débat sur les conclusions du rapport compétitivité une urgence pour redresser la ferme France. À la demande de la commission des affaires économiques. Je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire, Monsieur le Ministre de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour 2 minutes et l'orateur disposera à son tour d'un droit d'répartis pour une minute. La parole et tout d'abord aux orateurs de la commission des affaires économiques qui a demandé ce débat et monsieur Pierre. Au nom de la commission des affaires économiques pour 4 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre de l'agriculture. Et aussi Ministre de la souveraineté alimentaire et fait aujourd'hui qu'. On va vous le rappeler. Madame la présidente de commission, mes chers collègues. Le rapport que nous avons conduit avec mes collègues, Laurent Duplomb et Serge mais Riou expose à partir de cinq produits la pomme tomate blé les et poulet. Les raisons de la perte de souveraineté alimentaire de notre pays et propose à certaines solutions. Mais je comparerai la situation de l'agriculture à celle du nucléaire français. À force de maudire un système à force de maudire une façon de produire en faisant des règles en votant des lois doctrinaire et non réaliste le glissement vers une impasse était inexorable. En 20 ans, nous sommes passés du 2ème rang mondial des exportateurs à un déficit de production si on excepte les vins et spiritueux. Les agriculteurs baissent les bras comme EDF le fait depuis 10 ans. Nous avons beaucoup discuté ces dernières semaines de souveraineté énergétique, elle est indispensable mais tout indispensable et peut être encore plus et la puissance agricole d'un pays qui plus est un pays longtemps qualifié de grenier de l'Europe. Je remercie à ce titre. La commission des affaires économiques et sa présidente Sophie Primas d'avoir voulu inscrire à l'ordre du jour, un débat sur les conclusions de notre rapport sur la compétitivité de la ferme France rapport transpartisan et qui une fois encore tire la sonnette d'alarme sur la compétitivité de notre agriculture sur sa capacité à exporter ses productions comme à nourrir sa propre. Population. Les constats de ce rapport ne font hélas pas dans l'originalité puisque cela fait maintenant. Une vingtaine d'années que le Sénat alerte sur la perte descendante qu'empruntent notre agriculture. En 2015 déjà notre nous discutions d'une proposition de loi de notre ancien collègue Jean-Claude Lenoir sur la compétitivité de l'agriculture française. Pourtant chaque année qui passe, contribue à aggraver les déséquilibres maintes fois identifié fit bien que monsieur le ministre, il devient maintenant un périlleux d'agir. Notre rapport a mis en avant un certain nombre de facteurs contribuant à éroder voire à miner la compétitivité de notre modèle. Français, parmi ces 4 facteurs. Je voudrais en citer de la hausse des charges des producteurs en raison des coûts de main-d'oeuvre des surtranspositions ou encore d'une fiscalité trop lourde. Mais aussi une productivité en berne en raison d'un manque d'investissements, principalement dans l'agroalimentaire et dans l'élevage pour des raisons que nous connaissons, ici au Sénat que trop bien. Résultat, nos exportations. Implose. Et nos paysans désespère près d'un tiers de nos légumes sont importés. Les 2 tiers de nos fruits le son. Et que dire du poulet, dont près de un sur 2 qui est consommée dans notre pays n'est pas français n'étant plus capable d'offrir à nos compatriotes des produits agricoles de grande consommation accessible à tous. Face à ces constats alarmants nos recommandations n'ont pas vocation à rester lettre morte. Et je crois, Monsieur le Ministre que vous partagez nombre des constats mais aussi nombre de solutions préconisées dans ce rapport travaillant à leur ensemble à inverser cette tendance mortifère pour nos agriculteurs notre compétitivité, nos concitoyens et notre pays. Quand. Vous engage vous avec le Sénat, la vigilance la plus absolue quant aux surtransposition et ici je ne peux pas ne pas penser aux betteraviers, qui les premiers en Europe et au monde ont dû se passer des produits indispensables à l'état actuel des connaissances et de la recherche. Quand allez-vous pérenniser pour de bon les TODE pour sauver la filière fruits et légumes. C'était cher collègue je conclus je sais compter sur vous Monsieur le Ministre pour avec nous inverser cette tendance.

Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame, madame la présidente. Merci d'abord d'avoir organisé ce débat, ça permet de prolonger le travail qui a été fait. Et le rapport qui a été fait, qui pose des sujets comme ils viennent d'être évoqués par le sénateur lourd. D'abord vous avez raison, le sujet de la souveraineté, c'est un sujet qui traverse. Nos pensées, si je peux dire et nos actions politiques et la crise Covid, la guerre en Ukraine et un certain nombre d'événements viennent le le révéler plus encore pour ceux qui l'avait oublié. Crise énergétique, et autres sujets évidemment la souveraineté alimentaire est un élément très important. Je dis juste quelques mots et je répondrai à d'autres sujets, au passage, ça me permettra de répondre à vos questions Il me semble que la question de la souveraineté doit être posée à la fois au niveau européen et au niveau national, premier élément 2ème élément vous évoquez dans un certain nombre de sujets, la question de la capacité d'exportation de notre pays, c'est à la fois la capacité à subvenir aux besoins de notre population déjà et deuxièmement à reconquérir ce qui est notre place d'exportateur. Deuxièmement, vous évoquez la hausse des charges. Ou la hausse des charges globalement qui sont la question de la main d'oeuvre, ils ne sont que sur le CO2, même si on n'est pas complètement abouti, on a quand même fait un pas. De moyen terme avant d'être dans, sur un pas plus de plus long terme qui permet de donner un peu plus de visibilité 2ème élément sur la question de la fiscalité le qu'il faut qu'on et ce sera sans doute l'objet de la, du projet de loi d'orientation d'avenir sur la culture de repenser globalement la fiscalité à l'aune de ce que sont les besoins des agriculteurs. ce que sont les orientations qu'on veut donner et puis 3ème, élément de réponse sur la question des normes. Oui il y a une propension française qui n'est pas nouvelle. Un génie français. Je n'ose pas le dire mais qui est à, à celui de normer quand on a un problème et assure. Quand d'autres ont déjà. Vous avez raison de dire qu'il faut qu'on soit collectivement vigilants parce que ça nous a parfois échappé au cours des années. Il y a les normes européennes. Moi, dès lors qu'on est dans un cadre européen. Je peux comprendre, après il y a la question aux frontières mais dès lors qu'on est dans un cadre européen parce que beaucoup de la concurrence qui est exercée dans notre pays, c'est une concurrence à l'intérieur de nos frontières, par exemple sur les volailles d'ailleurs en partie sur les volets et donc on a besoin de se poser la question à chaque fois qu'on réglemente. Ou qu'on légifère juste poser la question de normes qui soit pas des freins à la compétitivité de la ferme France. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à monsieur Serge mais Riou au nom de la commission des affaires économiques pour 4 minutes. Monsieur le président. Madame la présidente. Monsieur le Ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Madame la présidente de la commission. Mes chers collègues. Pierre là dit avoir moi la situation de l'agriculture française est préoccupante. À bien des égards comme a montrer notre rapport de septembre 2022. je voudrais illustrer cette situation en vous parlant des éleveurs laitiers. J'ai pris. Un exemple, sur les cinq filières qui ont été étudiés dans ce rapport pour démontrer l'étendue de la crise dans laquelle se trouvent nos agriculteurs. 61% des éleveurs laitiers n'a terre d'atteignent pas le salaire médian. Monsieur le Ministre. 61%. Un agriculteur sur 2 partant à la retraite dans cette filière n'est pas remplacé avec comme résultante une décapitalisation du cheptel entamée dès 2005 et qui se poursuit inexorablement. Pourtant les prix du lait payé aux producteurs ont augmenté, plus 40% en moyenne sur un an dans l'Union européenne avec des sommets comme un Allemagne a plus 46%. Quant au prix moyen payé aux paysans français il n'a augmenté que de 22, 102 fois moins avec des charges qui elle aussi se sont considérablement accrues, comme vous le savez, comme toujours, l'agriculteur français l'éleveur et celui qui a le plus des difficultés à capter la valeur et manifestement Egalim n'a pas apporté les résultats escomptés. Alors, il est urgent, Monsieur le Ministre d'agir pour restaurer la compétitivité de ce que nous qualifions d'un autre rapport de miracle laitiers français tant le modèle familial de la ferme laitière française, qui nous est si cher paraît fragile face aux concurrents européens pratiquant une agriculture toujours plus intensive. Je rappelle que la France est désormais le quatrième importateur mondial de lait quand l'Allemagne bâti sa compétitivité sur ses performances techniques la France le fait sur la faiblesse de la rémunération de sa Ben-Dov Harmid familiale. Pourtant la France est aussi une puissance exportatrice. Mais elle a besoin d'un réel soutien de l'État. Pour aller conquérir ou reconquérir les marchés tout en protégeant le sien dans le cadre de nos travaux autour du rapport, nous ne sommes rendus en Italie pour voir comment on faisait au par-delà les Alpes. Hé bien Italie on assiste à une vraie promotion de leurs produits agricoles à l'international. Quel français n'a pas un été un morceau de mozzarella ou un peu de parmesan ne sort Peut-être même qui cuisine ça mozzarella avec des tomates italiennes mais croyez-vous que les Italiens ont eux aussi du comté ou de l'atome dans leur frigo cette promotion des produits italiens à l'international ne se fait pas uniquement sur des produits de haut de gamme pour s'en convaincre, il suffit de regarder les ventes de prosecco alcool festive et relativement bon marché en constante augmentation, alors qu'en est-il de notre stratégie à l'export de nos fleurons nationaux certes mais aussi de nos produits de coeur de gamme. Êtes-vous prêt Monsieur le Ministre, à travailler avec le Sénat a des solutions pour retrouver de la compétitivité de, de l'air à nos paysans soutenir la conquête de nouveaux marchés et surtout soutenir le marché français des produits venus du lointain. Ah l'aime pas qu'environnemental et social trop souvent catastrophique. Enfin à propos des denrées Bonnin, de loin, que pouvez-vous nous dire de cet énième accord de libre-échange de l'Union européenne cette fois-ci avec le Chili visiblement 5 clauses miroirs avec un pays utilisant des antibiotiques facteurs de croissance. Interdit depuis 2006 en Europe. Cet accord va-t-il dans le sens de l'histoire n'étant pas encore en train de sacrifier notre souveraineté alimentaire sur l'autel de notre souveraineté énergétique. J'ai cru comprendre que le sol du Chili était riches en métaux rares notamment du lithium bien utile pour nos batteries l'agriculture européenne et française est qu'une véritable qu'une variable d'ajustement d'accords internationaux aujourd'hui assez massivement rejetés par nos concitoyens. Parallèlement et par ailleurs je m'interroge sur le caractère peu démocratique de la manière dont la Commission européenne saucisson ne l'accord pour contourner les parlements nationaux. Je vous remercie. oui pardon. Merci monsieur le président, Monsieur Merieux, merci de vos mots alors je je j'ai répondu sur à la fois le lait et puis sur le, le dernier point, vous avez évoqué l'accord. D'accord sur le Chili et globalement les les accords internationaux mais j'y reviendrai j'imagine dans la soirée. D'abord sur les la question les tiers. C'est pas tant une question de souveraineté, à vrai dire c'est plutôt une question parce que sur le lait, on est plutôt. Alors en matière grasse, on est légèrement déficitaire mais en en matière protéique. On est Très puissamment excédentaire. La France est une grande puissance exportatrice les tiens. Ça ne m'amènera presque 2ème sujet mais je veux dire, il faut qu'on assume aussi la vocation qu'à la France et quand nos producteurs laitiers de faire en sorte que. On puisse. Participer de la balance du commerce extérieur d'un point de vue positif et de ce point de vue là, les données sont suffisamment rares d'un point de vue positif pour ne pas les soutenir 2ème élément. Vous avez posé le sujet qui n'est pas un sujet tant de souveraineté qui le sujet de la rémunération de la filière. De l'amont. C'est ce qu'on a essayé de mettre en oeuvre dans le cadre des Gallimard et des dégâts de je n'ai jamais dit que c'était parfait mes prédécesseurs non plus mais je pense qu'on a quand même avancé il y a eu un effet retard sur la filière et les rattrapages que vous évoquez, en particulier dans d'autres pays rupins sont en train de s'opérer en France qu'on savait qu'il y a un ou 2 opérateurs qui avait tardé à part à pratiquer Léo. Ce que nous avons désormais nous sommes déjà au mois de février mais ça a pu se faire récemment et je pense que c'est de nature à rassurer 3ème élément le risque principal, vous l'avez évoqué dans la filière laitière compte tenu d'ailleurs de la pénibilité du travail. C'est une activité qui mobilise 365 jours par an, matin midi parfois et soir sûrement, et donc il y a une question de travailler. C'est ce qu'on travaillera aussi ensemble je pense ou avec le Sénat, de travailler sur les conditions de travail la facilitation du d'exercice du métier de producteur laitier parce que le risque principal. Vous avez raison c'est tarif de décapitalisation. Et à terme donc de souveraineté et donc c'est là-dessus qu'il faut travailler encore. Enfin un mot sur l'accord du Chili, d'abord vous dire que. Il n'est pas en tout cas pour moi ni pour le gouvernement, la volonté de faire de l'agriculture une variable d'ajustement. La question c'est d'essayer de reconquérir des marchés. Vous avez-vous évoqué la vocation exportatrice de la France, on ne peut pas à la fois dire et on a une vocation exportatrice et je veux dire il ne faut pas qu'on dialogue dans la cave des accords internationaux. Le sujet principal pour moi c'est les clause de réciprocité les clauses miroirs qu'on a essayé d'introduire sous présidence française. Pardon je déborde un peu mais sous présidence française. Et qu'on doit encore cranter parce qu'on on a commencé à évoquer le sujet mais je pense qu'il faut qu'on aille plus loin pour qu'à chaque accord on puisse donner des clauses de réciprocité, ça c'est vrai. Merci monsieur le ministre. Monsieur Fabien Gay. Pour le groupe communiste. CRCE pardon.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente. Mes chers collègues. En ce début d'année, les syndicats paysans sont unanimes. L'inquiétude est grande avec une préoccupation majeure. Difficile de savoir si nos agricultrices et agriculteurs pourront vivre de leur travail en 2023. Les crises récentes nous ont montré l'importance de protéger nos filières du tout dérégulé. Déjà en 2021 pendant la crise Covid les intrants agricoles ont connu les plus fortes hausses de la décennie. Plus 10% sur les engrais, l'énergie, les lubrifiants, plus 11% pour l'alimentation des animaux. Il y avait certes tout un contexte, une pression sur les marchés des stocks approvisionnement limité des récoltes de céréales amoindrie par les aléas climatiques, les sécheresses le gel mais il y a aussi une inflation artificielle sur le marché de l'énergie qui vient de la spéculation sur les marchés boursiers, on le voit depuis l'agression de l'Ukraine par la Russie en plus d'une crise de l'approvisionnement. Il y a des profiteurs de crise, il y a du Trading et c'est un poste de dépenses qui a augmenté de plus de 370% entre 2021 et janvier 2022. Parce que là encore c'était marchés financiers qui impose les lois la spéculation à des hommes et des femmes qui veulent vivre de leur travail. Et ce système le gouvernement le cautionne. Vous avez refusé de rétablir les tarifs réglementés de vente pour toutes les. TPE et PME dont les exploitations agricoles et on s'étonne d'avoir une filière qui se demande si elle passera l'année. Quant au plafonnement à 280 euros le mégawattheure. Je pense qu'il faut être sérieux un instant, quand on passe de 42 euros le mégawattheure en 2021 à 280 euros en 2023. Il y a de quoi vous faire mettre la clé sous la porte. Alors Monsieur le Ministre, vous nous présenterez cette année une loi d'orientation et d'avenir agricole les agriculteurs et agricultrices vous attendront sur toutes ces questions comme sur votre politique commerciale. En l'espace d'un an de traités de libre-échange supplémentaires ont été conclus. Avec le Chili, mon collègue vient de le dire et l'autre avec la Nouvelle-Zélande. Donc moi je veux bien qu'on fasse une séquence émotion sur le recul de la filière bovine en France. Mais rien qu'avec ses deux traiter ces 12.000 tonnes de viande bovine qui s'est introduit sur le marché européen dopé à des substances interdites dans l'Union européenne. Et après il faudra dire à nos agriculteurs, il va falloir monter en gamme si l'on c'est fini c'est la retraite anticipée enfin si vous leur en laisser une parce qu'avec votre projet de réforme, c'est plutôt le chômage à 50 ans qui les attend votre projet d'agriculture, ce n'est pas celui du groupe communiste. Vous l'aurez compris, mais on peut avoir du débat et pour ça il ne faut pas, dans un propos en demi-teinte. Il faut assumer que vous défendez des importations venues de l'autre bout du monde qui font subir une concurrence déloyale à la filière française et aux filières européenne il faut assumer devant la jeunesse du pays qui s'est mobilisé pour le climat que vous signez pour des produits qui font le tour du monde, 20.000 kilomètres pour arriver dans nos assiettes, des produits qu'on sait faire ici. En meilleure qualité et ce n'est pas le simple fait des politiques européennes face auquel la France serait aussi impuissante pour ce traité avec la Nouvelle-Zélande. C'est la France qui avait la présidence de l'Union européenne, c'est la France qui s'est empressé de ratifier l'accord. Trois semaines avant la fin du mandat du président Macron désaccord nouvelle Gerardo génération comme on les appelle anti démocratique. En réalité, pour lesquels le Parlement n'est même pas associer d'ailleurs même pour les accords mixtes. On voit bien que vous n'avez pas envie de débattre. Il y a bien eu ici Monsieur le Ministre, vous le savez une résolution adoptée à l'unanimité pour que le CETA soit inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Cela fait 7 ans que l'Assemblée l'adopté à l'époque l'été qu'une simple Auchan enregistrement. Pour le gouvernement et toujours rien au Sénat par contre 90% du sept à s'applique aujourd'hui sur notre économie et sur notre agriculture s'étend d'application sans un vote sans bilan sans recul sans rien et la Dares la fois qu'un ministre, il m'a dit je vais vous emmener dans une exploitation agricole et vous verrez. J'attends encore c'était Monsieur Richter mais je vous refais la proposition si vous trouvez une seule exploitation pour lequel c'est bon je viens avec vous, sans caméra et je veux bien y passer une journée enfin les agriculteurs et les agricultrices mérite mieux que ce mépris et les temps que le débat ait lieu sur votre véritables politiques commerciales. Voilà je vous remercie.

D'abord. Il faut différencier. Vous parliez de la loi d'orientation et d'avenir. Il faut différencier ce que sont les sujets conjoncturelle de ce que ce sont des sujets structurels. Sur les sujets énergétiques la question si on est sur le structurel et le moyen et long terme c'est vrai récupérer si je peux dire de la souveraineté, y compris en termes énergétiques, c'est d'éviter de dépendre des autres, c'est un chemin qui est long c'est ça de, du 1er choc pétrolier, je pense que ça fait 50 ans qu'un certain nombre de responsables publics ont dit qu'il fallait qu'on sorte de la dépendance au pétrole. Donc ça va vite pour moi en tout cas à la modestie, mais en tout cas il faut qu'on essaie d'aller vers ce chemin là pour faire en sorte que on puisse. Pourvoir nous-mêmes à nos besoins énergétiques, c'est l'objet d'autres débats, y compris dans cette assemblée, mais je pense que c'est important de se le dire et c'est la transition vers des énergies moins carbonées et on le sait très bien, vous et moi, et puis deuxièmement, c'est un certain nombre d'éléments qu'on a mis sur la table. Je sais que les dispositifs sont pas tous parfaits pour essayer d'amoindrir le choc énergétique telles que nous connaissons je voudrais juste dire un mot des accords commerciaux. Ah vous dites faut assumer comme vous savez j'essaie d'assumer un peu les choses, y compris devant vous et je l'ai fait déjà devant votre commission. J'assume l'export et j'assume la vocation exportatrice de la France pour la filière porcine pour la filière laitière pour la filière vient et spiritueux pour la filière céréales c'est pas des petites filières tout ça. Et donc si j'assume l'export, j'assume les échanges et donc j'assume aussi dans parce que sinon c'est un jeu qui ne fonctionne pas les règles du jeu ne sont pas les bonnes. Si jamais on dit qu'on accepte de pouvoir vendre aux autres mais qu'on accepte qu'aucun produit ne viennent chez nous et donc on a 2 sujets le 1er sujet vous lever qui est assez juste ça c'est plus tellement le ministre de l'Agriculture. Seulement c'est le sujet démocratique. On a besoin au niveau européen de trouver des règles et au niveau national mais c'est Léon. Le gouvernement français ne fait que respecter les règles du qui sont fixés dans les accords internationaux de ce point de vue là, de trouver des règles qui permettent en transparence de dire les les accords les avantages des accords et puis 2ème élément je réponds juste sur la question du CETA. Paris tenu je vous emmènerai dans des exploitations, en particulier dans des exploitations laitières parce que le bilan du sept à aujourd'hui c'est 0 importations de viande bovine. Et c'est plein d'exportation vers le Canada de produits laitiers et donc je vous donne rendez-vous et on ira ensemble dans une exploitation laitière, y compris sans caméra. Merci Monsieur le Ministre, Monsieur.

Depuis quand. La nuit des temps l'Antiquité. Non mais je veux dire on a bien cours Marcé bien avant qu'on mette en place les traités de libre-échange libéraux. Au moins disant social et environnemental. Nous ce qu'on demande. Personne ne n'invite la France à se replier sur lui-même. On veut commercer avec d'autres. Mais avec les mêmes règles du jeu. C'est tout ce qu'on vous dit. Et donc vous avez un débat, c'est que ce que nous n'acceptons pas pour notre alimentation nos agriculteurs à nos agricultrices on les avec des produits qui font 4 fois le tour du monde. Et puis dernière chose, j'accepte de venir avec vous attention vous êtes le 3ème à me le dire. Julien Denormandie Franck Riester. Les 2 premiers ont pas tenu leur parole. J'espère que vous vous la tiendrai je vous remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente, chers collègues. Depuis près de 20 ans. Plusieurs rapports mettent en exergue la dégradation de la compétitivité de notre agriculture à de nos industries de transformation. Le rapport dont il est question aujourd'hui dresse à nouveau ce constat alarmant sur la situation, évolution qui pourrait conduire cela été dit d'ici quelques années à un déficit commercial agricole en 20 ans, la France est passée de 2ème à 5ème exportateur mondial en parallèle les produits importés ont doublé jusqu'à représenter la moitié de nos assiettes. Chaque jour la détresse de nos agriculteurs de nos exploitants et de l'ensemble des acteurs du monde agricole se fait entendre, et s'amplifie. Cela été dit en effet la question agricole est cruciale, particulièrement dans un contexte géopolitique troublé puisqu'elle porte sur notre souveraineté alimentaire notre capacité à produire notre propre nourriture aux conditions que nous choisissons, en toute autonomie, la compétitivité de la ferme France est mise à mal par 3 facteurs. Un coût de la main-d'oeuvre plus élevé que celui de nos concurrents pour exemple le coût horaire français a augmenté de plus de 50% entre 2000 et 2020, presque 2 fois plus rapidement qu'en Allemagne. Une surtransposition des normes qui accentue les distorsions de concurrence. Pour rappel, l'Union européenne autorise 454 substances actives au niveau agricole, mais au niveau national. La France n'en autorise que 309 enfin cette fameuse stratégie haut de gamme consistant à atteindre des marchés de niche plus rémunérateurs stratégie qui, il faut le dire. Produit de nombreux effets dévastateurs, notamment une baisse de notre potentiel productif, une orientation vers des produits plus honorer devenant inaccessible à de nombreux Français, cela nous conduit aujourd'hui à une perte sur le marché des produits coeur de gamme et au développement des importations pour faire face à la demande un non-sens dégringolade est revenu non respect des accords de libre-échange garder prix mitage des Terres agricoles, je m'arrêterai là sur le constat et pourtant Monsieur le Ministre, nous sommes une nouvelle fois sonné par l'inexistence d'un sursaut, d'un changement de braquet. Comme je le rappelais le 6 octobre dernier dans une question vous étant adressée, Monsieur le Ministre, mais rester malheureusement sans réponse satisfaisante les difficultés de la filière endives illustre parfaitement les problématiques de notre agriculture, baisse des prix. Pénurie de main d'oeuvre dans certains bassins hausse des coûts d'emballage et des besoins en eau ce secteur comme d'autres voix sa compétitivité se dégrader face à une concurrence toujours plus forte. Une concurrence ne s'embarrassant pas du pénalisant carcan normatif que nous imposons à nos agriculteurs, avec les membres de notre groupe Union centriste, mais plus largement, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme à l'occasion de l'examen des crédits agriculture lors du dernier projet de loi de finances. Les réponses n'ont pas été à la hauteur un. Une méthode et des moyens. Voilà ce qu'il est urgent de fixer aujourd'hui un cap qui doit reposer sur 3 priorités très claires, premièrement, nous devons faire de la compétitivité prix de notre agriculture une priorité nationale. Cela passera je passerais rapidement là-dessus cela été dit très concrètement par la mise en oeuvre une politique ambitieuse de réduction du prix du coup pardon de la main d'oeuvre en s'appuyant notamment sur une baisse des charges sociales par la montée en charge du dispositif TODE. Deuxièmement, je vous rappelle que notre agriculture est la plus propres du monde, il faut en faire un atout compétitif relance notre modèle agricole en dopant nos investissements et faisons de la ferme France une référence mondiale dans le domaine. Agricole nous devons stopper la multiplication des charges et des normes pesant sur notre agriculture Agriculture nous devons également garantir un principe pas d'interdictions de substances actives sans alternative et sans accompagnement. La filière betteravière en subit les conséquences aujourd'hui enfin utilisons mieux la marque France dans de nombreux secteurs à l'image de la viticulture, nous bénéficions d'une compétitivité hors prix inégalé en raison du prestige de la marque France et de sa crédibilité qualitatif pour finir Monsieur le Ministre, je formulerai un celui d'agir maintenant ensemble avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Merci cher collègue. J'ai le ministre. Merci monsieur le président, madame la sénatrice. M'avait dit un cap. Une méthode et des moyens. le quatre c'est celui que nous devons nous fixer de prendre conscience de la nécessité de la souveraineté c'est ça le cap, c'est de reconquérir de la souveraineté. Parce que c'est, vous l'avez dit, c'est très bien d'ailleurs décrit dans le rapport. Qui est l'objet du débat, il est évident que ça n'est. Pas ces 5 dernières années, ça n'est pas ces 10 dernières années c'est pendant 25 ans quasiment qu'on a laissé compétitivité. La la la compétitivité pardon de la ferme France. Et donc j'ai. Une responsabilité collective d'essayer de redonner cette perspective en regardant d'ailleurs filière par filière, ce que nous pouvons faire. La méthode pour moi c'est une méthode de planification. Je pense que la seule méthode que nous ayons devant nous pour essayer de relever ce défi-là c'est de dire. Quels sont les sujets, les impasses phytosanitaires pour ne citer que cet exemple dans lesquels on on est et quelles sont les alternatives qu'on doit produire pour éviter d'être simplement enfin c'est une interdiction sans au fond c'est ça ce que j'appelle la méthode et c'est valable pour tous les sujets. La question du carbone. C'est une question de substitution sur un certain nombre de filières. La question de l'énergie. C'est une question de même nature et donc c'est comme ça qu'on y arrivera, c'est par la planification, c'est-à-dire que lucidement sache où on veut aller. Qu'on ne recule pas d'ailleurs devant les obstacles et qu'on dise, on a un obstacle. On essaie de surmonter par la planification et peut-être que pendant 25 ans, on a essayé de dévoyer les obstacles et à la fin on finit quand même par se retrouver face à un mur et c'est le mur qu'on a, y compris par exemple qui a été évoqué. Tout à l'heure par le sénateur sur la betterave et donc on a besoin de trouver des alternatives et le les moyens c'est les moyens qu'on doit développer à la fois au travers de la recherche. Moi je crois beaucoup à la question de la recherche et l'innovation parce que c'est par la recherche et l'innovation qu'on trouvera des alternatives ou des voix différentes. Et c'est comme ça que. Vous sortir de la guerre par la mécanisation. Un peu plus tard par les produits phytosanitaires, on a réussi à stabiliser notre agriculture à portée de la rémunération. 2ème élément. Pour être rapide, je dis juste un mot sur la question haut de gamme. Et autres gammes. Essayons je sais que c'est un peu le, l'objet du rapport je je je ne partage pas ce point de vue d'abord. Près d'un tiers des exploitations françaises sont sous la belle et signe de qualité. Et ces exploitations là. Elle trouve de la rémunération, donc l'idée n'est pas de dire, il en faut moins. donc, n'opposons pas les systèmes par pitié. Nous pesons pas les systèmes on a simplement besoin de couvrir les autres besoins. C'est-à-dire que non mais donc c'est pas, ne fait d'avoir fait monter en gamme qui fait qu'on ait perdu la souveraineté c'est qu'on se soit un peu délesté des autres besoins des gammes monstre mais donc c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille mais on a besoin d'AOP IGP GP de signes de qualité, vous en avez dans tous vos territoires. Je ne connais pas un producteur qui soit sous signe de qualité qu'il renoncerait aux signes de qualité pour faire d'autres gammes. Peut être sur le dernier point sur la montée en gamme. Je n'ai pas dit l'inverse de ce que vous dites. N'est pas contre, je dirais cette offre de monter en gamme mais ce qu'on est en train de dire c'est qu'en faisant ça on fait un choix et on oublie tout ce qui aujourd'hui n'ont pas accès à ces produits-là et donc forcément quand on fait un choix on renonce à d'autres. Donc là ce que je dis juste. Oui, sauf qu'on a fait un choix qui était peut-être démesuré aujourd'hui et qui fait qu'on laisse sur le bord de la route, un trop grand nombre de Français qui aujourd'hui n'arrive plus à consommer les produits produits en France, en France, c'est ce que je dis. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques. Mes chers collègues. Qualité vs quantité le rapport que nous examinons aujourd'hui opposerez ces 2 modèles. Je me refuse de rentrer dans ce débat, notre agriculture est plurielle conventionnel achever raisonnée bio il y a de la place pour tous. Mais j'adhère complètement au contexte qui a généré ce rapport, nous ne sommes plus compétitifs. C'est évident et ce n'est pas de maintenant. Nous avons tous notre part de responsabilité. Avec un constat, la ferme France s'affaiblit s'appauvrit les chiffres en attestent. 100.000 c'est le nombre d'exploitations perdu au cours des 10 dernières années. Avec un taux d'agriculteurs dans l'emploi passé de 7% en 1982 à 1,5%. Anne 2019. Quel jeune va choisir ce métier. Avec des prix non rémunérateur et des coûts exponentiels, a fortiori avec l'augmentation des matières premières qui sera tenté. Les agriculteurs sont les seuls qui ne décide pas du prix de leur production. On leur impose un prix, en faisant fi de tout le coût de leur production. Une affection qui s'ajoutent aux éléments exogènes qui subissent de plus en plus aléas économiques climatiques, sanitaires et dont on parle souvent dans cet hémicycle. Il subissent, c'est la volonté de la grande distribution, mais on peut agir en amont, les organisations professionnelles doivent avoir des Liens Directs avec les consommateurs, connaître l'évolution des goûts des besoins construire des stratégies s'adapter au marché est au minimum et pourtant certaines filières n'ont pas su le prendre. Nos voisins espagnols se sont structurés par secteur avec des stratégies collectives très efficace sur les marchés européens. En France on se concurrencent les désole des autres. Prenant l'exemple des coopératives viticoles que je connais bien nombreux en Occitanie. Sur un même territoire, on était incapables faire une offre globale hein produisant les mêmes 20 chacun pour soi. C'est une voie facile pour les scènes négocié négocié en face qui du coup joue la division in fine et il fixait les prix et rendent dépendants c'est pareil d'ailleurs pour d'autres filières. Il est urgent de fixer des enjeux nationaux des enjeux régionaux pour décider de stratégie commerciale et d'images efficiente car notre agriculture. C'est ce qui dans ce marché mondial où la concurrence est exacerbée. Mais nous, nous partons pas il est vrai à armes égales. Les charges sociales, les normes diffère et nous agriculteurs pâtissent de ces de ces inégalités. Dans le rapport, il est question de de lourdeurs administratives souvent cité par les les agriculteurs en difficulté les formulaires s'accumulent et prennent une large part du temps de travail. Là et lorsque l'on sait qu'ils travaillent plus de 60 heures par semaine la simplification vieux serpent de mer plus qu'acteur réel s'impose vraiment. Monsieur le Ministre vous défendez vos administrations et c'est évident. Mais les faits sont là, les dossiers aussi là. Le dernier pour lequel on m'a interpellé, date de la semaine dernière. Jeune agriculteur de 26 de 26 ans. Se voit refuser plus de 20.000 euros car il n'a pas donné un formulaire ou qu'il a oublié de cocher une case dans une demande de Pâques. Alors oui il peut perdre son entreprise et s'énerver. Le droit à l'erreur, devrait s'imposer là bien devrait s'imposer aussi. Cette lourdeur bien caractéristiques à la France participe à d'autres baisses de compétitivité. Sur le ministre, je vous invite à remplir un dossier pas. À compter les arbres par exemple de cocher les les les mêmes occase du parcellaire chaque année alors qu'on pourrait indiquer seulement ce qui a changé. Je l'ai vécu en Direct pendant plus de 8h. Une fonctionnaire de la DDTM de l'Hérault, très impliqué très humaine m'a aidé car il a fallu que constitue mon dossier par ceux d'air perdu par les services. Elle m'a expliqué que chaque pays membre à son propre logiciel en Italie d'où elle est originaire. Il est bien plus simple. Pourquoi, pourquoi c'est plus sympa d'Italie. Que vous le nom réellement les solutions existent, certaines dans le rapport. Stop surtransposition augmenter les crédits à l'innovation et à la recherche, développer les contrer les les contrôles. Un exemple de la loi Egalim a imposé à la restauration collective 50% de produits de qualité, durable, donc 20% de bio qui l'année le bilan. La stratégie doit être globale. Quelle vision pour notre agriculture, quels enjeux. Avec quels moyens. Lorsque nous avons proposé avec ma collègue Françoise Férat, de placer l'agriculture à 2023 grande cause nationale comme premières préconisations d'un autre rapport sur le mal-être des agriculteurs. Ce n'était pas symbolique, c'est primordial. S'est montré un signe fort à nos paysans c'est passé le foncier agricole la formation les paiements pour services. Manteau l'eau la souveraineté alimentaire comme sujet fort étudier ensemble plus qu'autre plutôt que de travailler le sujet par sujet, Le coup par coup à l'efficacité les gens je les âges sont transversaux les solutions doivent l'être aussi. Je vous remercie, monsieur le président, Monsieur le Sénateur Cabanel vous avez-vous. Beaucoup de sujets, donc je vais essayer de répondre. Au moins deux minutes Monsieur le Président parce que j'ai débordé tout à l'heure, d'abord pour vous dire vous avez évoqué la sujet. De la rémunération, c'est ce à quoi on essaie de répondre au travers des gamines, je ne dis pas, je le répète que c'est parfait, il y a vous, À examiner un texte qui vient aussi compléter un certain nombre de dispositions mais je pense qu'on va dans le bon sens et je ne connais personne d'ailleurs, qui disent que ça n'a pas été dans le bon sens sans égaler mais quand je crois d'ailleurs d'autres collègues européens. Et pas qu'européen. Compris les Canadiens me disent on est intéressé par ce que vous faites par Egalim parce que vous construisez le prix par le coût de production et par la matière première et par l'amont et non par Laval. Et on a besoin aussi dans le dialogue qu'on a avec nos concitoyens de ne pas se laisser embarquer sur inflation versus rémunération. Parce que depuis 45 ans ou de 50 ans ou un peu plus, on nous explique que ceux qui défendent la lutte contre l'inflation. C'est ça, c'est une cause nationale qui défendent et ça se fait généralement sur le dos des agriculteurs. Parce que ça a un coût, ça a un prix. Il faut qu'on le dise et parce qu'on a des exigences environnementales qui sont particulières chez nous et qu'on a des exigences tout court ça ça a un coût et donc ça a un prix et donc il faut aussi mener ce combat-là parce que sinon on mène pas bien le combat. Le combat de la juste rémunération est un combat et qui est encore devant nous et pas se laisser embarquer sur la question de l'inflation 2ème élément. Vous avez raison, on a besoin de coopération entre les filières et et à l'intérieur des filières. Parfois je regrette moi-même qu'on puisse pas mieux coopérer parce que ça n'est jamais les filières qui ont prévu bénéficient de cette absence de coopération, c'est les tiers qui tirant parti des divisions et c'est d'en tirer le meilleur parti pour eux en terme de rémunération et de prix 3ème élément le droit à l'erreur. Je sais que vous m'avez saisi du dossier particulier mais vous avez raison, on a besoin je ne dépends pas les administrations sûrement par principe parce qu'elles font d'abord. C'est la responsabilité du législateur de celui qui fait le règlement et du gouvernement et donc je prends ma part de responsabilité. ça serait se défausser de dire que c'est de la faute des administrations c'est notre responsabilité collective et malheureusement c'est un peu le génie français entre guillemets. Au mot génie qui fait que, à chaque problème nous étions crée une réglementation et c'est vrai que la qu'à la PAC française telle qu'elle est posée, elle est beaucoup plus compliqué chez nous que dans d'autres pays tiers mais c'est je crois qu'on l'a fait parce qu'on a voulu tenir compte de telle ou telle différence de telle ou telle attente de telle ou telle demande de telle ou telle de telle ou telle climat enfin bref on a créé un système complexe au passé qu'après l'administration soit mais on a besoin du travailler et d'avoir une forme de bienveillance parce que, y compris dans la PAC qui c'est en train de se se déployer en 2023 on a besoin sur des systèmes nouveaux de l'expliquer mieux hé bien pour que les agriculteurs ne soient pas pris en défaut de ce qui est quelque chose qui relève de la bonne foi. Alors pour eux si si si si un petit peu de temps mais vous avez débordé donc. Merci. Merci monsieur le prix de, je ne savais pas long. Vous avez bien compris l'interrogation qui est celle de l'agriculture d'un et je veux insister sur la complexification de l'administration. L'administration est là pour nous contrôler et je pense que les agriculteurs l'acceptent. Mais elle est elle est là aussi pour nous aider. Et quand on voit donc le désespoir d'un certain agriculteurs. je l'ai dit dans. Mes propos mais j'ai insisté, vous l'avez aussi évoqué. On a besoin de bienveillance et là vos organisations dans les administrations, la, la Mutualité sociale agricole. On a besoin de bienveillance et les agriculteurs, ce ne sont pas simplement des chiffres de la Mutualité sociale agricole. C'est des femmes et c'est des.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'agriculture est une chance formidable pour la France. La crise de la Covid 19, a rappelé l'importance stratégique de l'agriculture et des agriculteurs qui se sont engagés, tout au long de cet épisode sanitaire. Pour nourrir les Français alors qu'une partie du pays étaient à l'arrêt. À l'heure où l'équilibre du monde, est déstabilisé par le conflit russo-ukrainien la souveraineté alimentaire n'est désormais plus une option, mais une nécessité pour la France qui a été et doit redevenir une grande nation agricole. Néanmoins, pour réaliser cet objectif, il est indispensable de jeter un regard critique sur l'ensemble de notre politique agricole de la production jusqu'. Au consommateur final. C'est tout l'objet du rapport d'information de la commission des affaires des affaires économiques réalisés par nos quatre collègues rapporteurs dont je salue ici le travail. En effet, comment ne pas s'inquiéter lorsque l'on observe que la France se trouve être l'un des seuls grands pays agricoles, dont les parts de marché recul passant de la 2ème à la 5ème place d'exportateur mondial en 20 ans. Dans un même temps et comme le souligne le rapport. Les importations alimentaires en France ont doublé depuis 2000 et représente parfois plus de la moitié des denrées consommées par les Français. Il en va de même pour la viande bovine en Net recul. La France a perdu 11% de son cheptel en six ans seulement, soit 837.000 vaches et mon département de la Mayenne n'est pas épargnée. En 10 ans. On est passé de 600.000 bovins à 530.000. Cette situation est particulièrement inquiétante au regard des importations de viande bovine quant à elle, qui ont augmenté de plus 15% sur un an. Entre 2021 et 2022, un quart du boeuf consommé en France est importé, contre moins de 20%. Quelques années plus tôt. Bien sûr, comme le souligne également le rapport de nombreux facteurs entrent en jeu pour expliquer cette situation. Le non-renouvellement générationnel des agriculteurs et problématique entre 1982 et 2019 le nombre d'agriculteurs a été divisée par 4 passant de 1,6 millions d'agriculteurs à 400.000. Le constat étant dressé, il nous faut désormais mettre sur la table et solutions qui permettront de redresser la ferme France et de préserver notre titre de puissance agricole. Il nous faut pour cela crée un choc de compétitivité qui passe d'abord par l'aîné CERS c'est la nécessaire simplification des normes applicables aux agriculteurs. Il est indispensable de donner aux agriculteurs de la clarté de la visibilité sur des normes sanitaires, environnementales administratives qui ne cessent d'évoluer. Pour ne citer qu'un exemple récent, l'Union européenne est en train de se pencher sur une révision des normes de commercialisation visant à changer les règles d'étiquetage des modes d'élevage des volailles ce qui menace désormais la production de volaille fermière particulièrement implanté dans l'ouest de la France. Pendant ce temps nos accords de libre-échange autorise l'importation de denrées alimentaires dont les normes de production sont loin des standards européens avec un coût logiquement réduit. Nous sommes donc d'un côté en train d'asphyxier nos agriculteurs sous des normes et des surtranspositions que nous n'exigeons pas des pays hors Union européenne. D'un autre côté, nous créons de France, une France qui peut s'offrir des produits européens plus cher en raison des normes et une France qui achètent et consomment des denrées importées qui échappe à certains contrôles. Cela doit cesser. Il nous faut aussi d'urgence engagé un choc de simplification pour notre agriculture, et une révision des accords de libre-échange. Ces 2 conditions sont indispensables pour permettre à nos concitoyens de consommer français à un coût compétitif. Le défi du renouvellement générationnel auxquels est confronté notre monde agricole doit également faire l'objet d'une action urgente, il nous faut renforcer l'accompagnement des jeunes agriculteurs, notamment avec la dotation jeunes agriculteurs et les banques doivent également jouer jouer leur rôle en permettant de mettre à disposition des jeunes agriculteurs des interlocuteurs véritablement à l'écoute de leurs projets. Enfin le dernier chantier est incontestablement celui de l'adaptation de notre agriculture au réchauffement climatique. Que ce soit en matière d'utilisation de la ressource en eau. Que au niveau de la gestion des catastrophes naturelles. Il est indispensable de soutenir les agriculteurs qui investissent dans des équipements d'irrigation. Moins consommateurs en haut et plus performant. Convient aussi de mieux protéger. Nos exploitations agricoles dans le cadre du dispositif de catastrophes naturelles, comme bon nombre d'entre vous, on a pu constater des dégâts importants à la suite des grêles sur nos cultures en à, au, au printemps dernier d'ailleurs, Monsieur le Ministre, vous êtes venu dans mon département, il est de notre devoir d'accompagner de mieux soutenir ceux qui subissent ces pertes comme cela a été fait avec le système d'assurance-récolte réformer. En résumé, il nous faut nous donner les moyens de travailler avec nos agriculteurs une législation. Plus équilibré. Il y a des accords internationaux plus juste il y a donc du pain sur la planche, Monsieur le Ministre. Est ce que vous tenez sous les 2 minutes. Ça n'est pas un sujet. Europe versus sur le reste du monde, c'est un sujet européen c'est une demande un certain nombre d'États de l'Union européenne de, de réviser les normes de commercialisation. Donc nous sommes en train en européen à l'intérieur des frontières de l'Union européenne de faire en sorte que nous préservions. Au fond c'est presque, antinomique avec ce que je dis parfois dans le rapport, ce que nous préservions. Ce qui est une forme de la belle qui le Label plein air parce que c'est ça le sujet hein sur la volaille. Donc c'est pas un sujet de descente en gamme, c'est un sujet de monter en gamme et donc on veut défendre dans le modèle européen, notre spécificité parce que nous sommes le pays qui a le plus développé cette question de, de la volaille plein air on est en train d'essayer trouver un chemin, je ne peux pas vous en dire plus. Ça date, puisque nous sommes dans une phase de négociations, mais la volonté c'est bien de défendent le modèle sur lequel nous nous sommes appuyés pour développer un certain nombre d'élevages 2ème élément sur la question, je reviens sur les les accords de libre-échange dis je dis juste un mot. Général, il y a à la fois de faire en sorte d'assumer la capacité et la vocation exportatrice de notre pays que nous avons et que nous avons en partie perdu. Deuxièmement d'avoir des clause de réciprocité. Troisièmement je pense qu'on a besoin de travailler sur, quand vous regardez d'autres pays européens qui sont parfois avec aussi les mêmes contraintes. Normatives hein pour un certain nombre d'entre eux et je pense qu'on a besoin d'assumer une politique beaucoup plus offensive sur les marchés extérieurs. Je pense que pour le coup, là on aurait intérêt à regarder sur un certain nombre de marchés émergents ce que nous pouvons faire pour conquérir des marchés, enfin vous avez évoqué la question de l'installation des jeunes cidriculteurs, pardon de le dire un peu brutalement. Je ne suis pas sûr que la question du montant de la DGA soit le seul sujet d'abord. Plus de la moitié ou près de la moitié des jeunes qui s'installent ne bénéficient pas de la DGA. Donc on a un sujet de la cible. 2ème élément compte tenu des montants, y compris des montants de capitaux qu'il faut engager. Quel que soit le montant de la DGA on a besoin de de de de rassurer de réassurer le jeune agriculteur sur son revenu sur la capacité à rembourser des emprunts et sur la capacité, là vous avez raison, à faire face au dérèglement climatique, c'est plutôt autour de ça en particulier qu'il faut qu'on essaie de travailler, on a besoin de dans ce monde déréglé climatiquement géopolitiquement économiquement. De faire en sorte que le système où on puisse se dire qu'à 30 ans il tient c'est comme ça qu'on l'installera des jeunes agriculteurs. Merci Monsieur le Ministre, la parole est à monsieur Franck Menonville pour le groupe les indépendants pour cinq minutes.

Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre agriculture façonne le paysage français. Elle fait partie de notre ADN national elle est aussi la base de notre patrimoine culinaire avec ses fromages, ses cultures, ces viandes, c'est 20 ces terroirs et sa diversité. Mais le constat pour notre agriculture française devient préoccupant. Notre collègue Laurent Duplomb dans son rapport de 2019 mettait déjà en évidence le déclin de notre agriculture. Force est de constater que rien n'a changé. La crise actuelle a même renforcé certaines difficultés notamment dans l'élevage. Notre production stagne voire recule dans certains secteurs depuis 1990. Nous sommes le pays qui connaît la plus forte baisse de part de parts de marché depuis 2000, copain compétitivité s'effrite, nous perdons donc des parts de marché à l'export en parallèle nos importations progressent. Elles, elles ont plus que doublé en 20 ans et nous important aujourd'hui 63 milliards d'euros de denrées alimentaires. Pourtant notre agriculture dispose d'un potentiel incontestable en effet la France est le principal producteur européen, loin devant l'Italie et l'Allemagne. Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire d'une telle évolution. Il est urgent d'agir. je salue vraiment véritablement le travail de nos 3 rapporteurs qui pointent la baisse de compétitivité liée aux 4 constat effectué ce travail essentiel et pertinent met en avant en s'illustrant sur la réalité de cinq filières et fait 24 propositions. La période actuelle nous oblige à réaffirmer notre souveraineté alimentaire. Nous devons agir rapidement, car notre autonomie alimentaire est mise en péril. À titre personnel et ça a été évoqué par notre collègue. Madame Gacquerre. Je pense que la stratégie du monter en gamme prônée notamment par le président de la République dans son discours de Rungis ne peut définir à elle seule notre futur agricole. Nous devons être présents sur tous les créneaux toutes les gammes le haut de gamme. L'entrée des mais également l'entrée de gamme pour répondre aux attentes de tous les consommateurs. L'augmentation des importations sur certains produits et le recul du bio sont des signes plutôt clair, cette tendance s'est d'ailleurs accrue depuis. Cette crise Après la lecture du rapport, j'ai choisi de mettre en lumière un problème qui a été. Très bien identifié, celui des surtranspositions, trop nombreuses et des lois franco-françaises trop strict. À titre d'exemple, 454 substances actives sont autorisés au sein de l'Union européenne alors que la France n'en autorise que 309. Nous devons nous ne pouvons pas donc imposer des règles. nous pouvons pas imposer des règles que nos voisins ne s'impose pas eux-mêmes. Nous ne nous devons donc imposer à nos frontières et nous devons imposer à nos frontières. Ce que nous exigeons de nos agriculteurs. Nous devons donc poursuivre notre harmonisation européenne pour éviter la concurrence intra et extra-européenne qui nous pénalise c'est pour soi. Il me semble que la reconnu la recommandation numéro 2 de ce rapport est très intéressant pour donner donc corps au principe Stop aux surtransposition, grâce à la à une mission qui. Pour être donné donc au Conseil d'État. L'exemple de la filière betterave. Betteravière donc illustre bien ce sujet un arrêt donc de la Cour de justice européenne vient d'interdire la dérogation concernant les néonicotinoïdes. La filière est aujourd'hui dans une impasse technique pour lutter contre les pucerons verts et la jaunisse. Je rappelle que la France est le premier producteur de sucre de l'Union européenne cet exemple met en évidence une nouvelle fois la mise en péril de notre souveraineté par des législations mal adapté aux réalités de des territoires.

pour éviter donc toutes les impasses techniques. Qui fragilise durablement les filières. Monsieur le Ministre, nous connaissons votre engagement, vous êtes bien sûr pas comptable de cette situation dégradée. Il faut donner à nos agriculteurs les moyens de la performance et de la compétitivité et nous serons à vos côtés pour remplir cet objectif. Ne faisons pas de notre agriculture. Ce que nous avons fait de notre industrie. Il est urgent d'agir. Les agriculteurs français sont motivés, passionnés, ils aiment leur métier mais de les surcharge administrative et les complexités de nos politiques publiques freine l'attractivité de la profession. Il est important donc de leur redonner du sens et des perspectives pour que de nombreux jeunes. Veuillent s'investir et s'installer dans ce merveilleux métier. Monsieur le Ministre, comptez-vous comment comptez-vous donc utiliser les recommandations de ce rapport. Pour. Transpartisan comme base de travail pour l'élaboration un et de la loi agricole. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre. Hein. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Sénateur Menonville. Merci de vos questions. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à coeur comme à vous tous ce soir. Je vais le prendre dans l'ordre inverse d'abord la question des surtranspositions. Vous trouverez pas au moins. Ministre de la culture qui cherche d'être sur-transposition et qui les recherches. Oui on est un pays qui a tendance à, à penser que parce qu'il devrait être en figure de proue et d'avancer. Sur un certain nombre de sujets. Ça fait 25 ans que ça dure hein. On pense toujours qu'on est là, à dire on va le faire les premiers, les autres les suivront, sauf que généralement les autres nous regarde et que dans l'intervalle on a perdu en compétitivité ou en souveraineté ça veut dire qu'on a d'abord un sujet sur question de normative. À débattre au niveau européen. Quand c'est une décision, un choix qui est fait au niveau européen pour le coup, ça c'est des sujets. Que y compris nos agriculteurs peuvent comprendre sous la réserve que dans les accords commerciaux. On essaie de trouver des clause de réciprocité. Donc ça vous le trouverez toujours ce chemin-là on est aussi dans un cadre juridique, je vois bien que vous faites appel éventuellement au Conseil d'État. Le principe de précaution, le principe de régression. C'est pas ce gouvernement, c'est pas celui d'avant c'est pas celui d'avant c'est pas celui d'avant mais c'était il y a très longtemps, simplement, c'est dans la Constitution pour un certain nombre de ces éléments-là à penser que nous pourrions facilement oeuvrer en tout cas chaque fois qu'on peut avancer sur l'idée qu'on ne sur transpose pas et qu'on n'est pas forcément à penser qu'on est meilleur que les autres dans ces domaines-là parce qu'on on porteurs en avant les sujets et pour les au niveau européen. J'ai aucune difficulté avec sa 2ème élément sur les montants. Je suis d'accord avec vous, on a besoin.

de monter en gamme et la capacité de répondre, je prends juste la volaille. Oui on a besoin de redévelopper des élevages vol de volaille en France pour assurer simplement notre souveraineté et donc je l'assume très pleinement parce qu'on ne peut pas à la fois dire, on n'a pas de souveraineté on exporte au fond du carbone on exporte des pratiques dont on ne veut pas. Et on refuse en même temps de faire le moindre élevages de volailles sur notre territoire. Ça c'est pas possible parce que là il y a une contradiction et donc vous ne trouverez sur le chemin d'essayer de retrouver la souveraineté sur ce sujet là par exemple je donne l'exemple de la volage ce que ça faisait un exemple qui est effectivement parlera et puis dernier élément, Désolé. Bon. Répondrai tout à l'heure sur la marque France. Merci monsieur Daniel Salmon pour le groupe écologiste solidarité et territoires pour. Cinq minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, madame la présidente. Le rapporteur, mes chers collègues. La question de la compétitivité de la ferme France suppose de se mettent d'accord déjà sur la définition que l'on accorde à ce terme. Ainsi, pour le rapport dont nous débattons ce soir la compétitivité se défini via des prix des volumes et des coûts de production sur un marché. Internationaliser mais cette définition doit aussi nous interpeller. En effet la notion de compétitivité ne peut continuer d'occulter des dimensions multiples assumer de façon collective. Que devient notre compétitivité, si l'on intègre les coûts cachés des pesticides chiffrée entre 370 millions et plusieurs milliards d'euros par an pour la France, que devient-elle si on calcule les impacts des engrais azotés sur le climat, l'eau et les sols a-t-elle un sens si l'on oublie l'impact des pratiques agricoles sur les pollinisateurs et sur la fertilité des sols dont nos cultures dépendent. A-t-elle un sens sans analyser ses effets sur l'emploi ou la qualité nutritionnelle des aliments. On peut aussi évoquer pour questionner cette fameuse compétitivité. Les très fortes subventions publiques qui mettent sous perfusion perfusion le système agro-industriel. Rappelons que sur les 23,2 milliards d'euros de fonds publics versés chaque année à peine 1% a un effet sur la réduction de l'utilisation des pesticides. Certes, nous ne pouvons pas nous affranchir en un jour du marché mondial et de ses règles, mais nous pouvons agir pour mettre fin aux accords de libre-échange pour des clauses miroirs une régulation des marchés pour une relocalisation de notre alimentation. Alors que de plus en plus de citoyens sont en situation de précarité et sont contraints de baser leur choix alimentaires sur les seuls prix il est de notre responsabilité de garantir l'accès de toutes et tous à des produits sains et durables. Nous avons et ce qui s'est, d'épices dans le rapport de notre collègue Mélanie Vogel, sur la sécurité sociale, écologique dans une partie portait sur l'alimentation. Vous l'aurez compris, pour nous, la solution n'est pas de subventionner encore et toujours plus la supposée compétitivité d'un modèle agro-industriel à bout de souffle. Il nous faut, au contraire, construire une véritable compétitivité intégrant toutes les externalités positives ou négatives de nos systèmes agricoles. Je voudrais ici insister sur un modèle agricole qui répond à cette notion de performance globale à la fois en termes de production, d'emploi, de respect de l'environnement de santé publique et de relocalisation. Il s'agit. Cela ne vous surprendra pas de l'agriculture biologique. Ce mode de production qui connaît des difficultés reste pourtant plus que jamais compétitifs, c'est une production locale consommées en majeure partie localement elle stocke l'eau dans les sols. À un moment où on en a besoin à l'heure où nous connaissons des sécheresses de plus en plus intenses en respectant la saisonnalité et les vitres de chauffage des serres à l'heure où l'explosion du prix. À l'heure de l'explosion du prix de l'énergie. Elle se passe des engrais azotés, dont le coût a flambé et donc moins touchés par l'inflation et par les aléas géopolitiques. Et pourtant, face à un ralentissement de la demande, il semble que le gouvernement. De laisser en difficulté ce modèle porteur de solutions d'avenir. Car ce sont bien des politiques publiques inadéquate qui nous conduisent à la situation actuelle. Je citerai ici la promotion de la HVE qui n'apporte pourtant aucune véritable garantie actant la confusion du message autour des atouts de la bio pour l'environnement et la santé. La fin de l'aide au maintien dans la nouvelle PAC et donc l'absence de rémunération des services éco-systémique de la bio. On peut aussi évoquer le soutien minimal de l'État aux opérateurs de la bio en particulier l'Agence Bio dans le rôle pour soutenir la demande est pourtant primordial. Je pourrais continuer car un rapport de la Cour des comptes détaille bien d'autres politiques qui n'ont cessé de pénaliser l'agriculture biologique. Ces dernières années et alors que ce ne sont ici que des exemples. 489 millions d'euros d'aide à l'achat pour l'alimentation animale ont été débloqués dans le cadre du plan de résilience, ainsi que 270 millions d'aide d'urgence ont été mises sur la table pour la filière porc conventionnelle depuis un an. Rien n'est fait pour soutenir la bio. Nous regardons donc des agriculteurs se des convertir ou arrêter leur activité des outils de transformation se perdre. Allons-nous demain du bio, car nous aurons laissé se déstructurer une filière entière. Nous souhaitons donc ce soir vous interpeller monsieur le Ministre, sur la mise en place d'un plan de soutien pour cette agriculture. Il est plus qu'urgent de déclencher tous les mécanismes pour aider la filière notamment des aides d'urgence à l'actif et un plan ambitieux de communication a minima une partie des financements destinés au développement de la bio comme les aides à la conversion ou le Fonds Avenir Bio pourraient être basculé sur l'aide aux entreprises et exploitations en difficulté dans l'attente de réponses plus structurelles des leviers multiple sont à la disposition du gouvernement. Nous attendons que vous les actionner. Allons nous mettre la tête dans le sable pendant 40 ans comme nous l'avons fait face au climat et ici face à l'effondrement de la biodiversité. Parce que cet effondrement est en cours. Et je pense qu'ici. Certains trouvent qu'il y a encore beaucoup trop d'insectes. Mais je n'ai pas mon cas. Merci cher collègue. Monsieur le Ministre. Merci monsieur le président. Merci monsieur le sénateur. Vous avez. Évoqué la compétitivité sous un regard qui est le qui est le vôtre, en vous écoutant, je me suis dit que. vais, j'espère ne pas être offensant que c'est comme ça qu'on s'est posé des questions sur le nucléaire et nous que nous retrouver dans les mêmes difficultés ont terminé gentille parce qu'on nous a expliqué que la solution. C'était pas le nucléaire c'était les énergies renouvelables sans nous donner le traître mot le moindre mot de la façon dont on y arriverait là vous nous dites, la solution c'est le bio et ça répond à toutes les questions. Pardon moi je n'ai pas envie de me retrouver dans les mêmes impasses de souveraineté, je vous le dis très clairement. On peut aussi tirer, exemple de ce qui s'est passé ces dernières années. Ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas besoin nécessité et envie de soutenir l'agriculture biologique mais par pitié, essayant de ne pas opposer les systèmes. Le bio, il a un problème qui est un problème de demande. Donc vous pouvez le faire comme vous voulez. Non mais pourrait le faire comme vous voulez mais si vous voulez pas vous confronter à la réalité du marché et que vous produisez quelque chose que les consommateurs ne prennent pas. Vous vous posez la question du segments de marché, donc on a besoin de travailler avec la filière bio, non pas à dire on produit en produit en produit c'est comment on arrive à ce que les consommateurs puissent s'intéresser à la filière. Parce que sinon on va dans le mur, on produit quelque chose que les gens ne consomment pas alors on peut vivre sur une île déserte et sur une théorie économique. Vous dites la compétitivité je la vis à mon échelle mais pardon. Quand bien même nous soyons insulaires. Nous vivons dans un monde où il faut nourrir les gens. Où il faut nourrir par-dessus, nos frontières parce que notre intérêt, c'est que quand même à nos frontières extra-européenne des gens trouve à s'alimenter donc. Pardon, on a besoin de de d'être dans le réel. Dans cette affaire-là et donc vous nous trouverez sur le chemin de soutenir la bio. Vous êtes un, un élu de la Bretagne. Vous proposez quoi de supprimer les aides qu'on a fait à la filière porcine vous ne supprimez vous proposez quoi de supprimer les aides qu'on a fait, qui était conjoncturel à l'alimentation qui a, qui ont concerné les bio et lait conventionnel. Tout le monde donc je veux dire je veux bien qu'on fasse toutes les ruptures qu'on veut mais il y a un moment il y a des réalités qui s'imposent et la réalité qu'on a, c'est à la fois d'assumer les transitions et je les assume parfaitement et en même temps vous de pas imposer un modèle unique parce que le modèle qui nous met dans une impasse. Je vous le garantis en termes de souveraineté. Si Monsieur le Ministre. Seulement. Monsieur le ministre je vous rappeler que la plus grande réalité c'est la biosphère. Et effectivement, je suis en Bretagne. En Ille-et-Vilaine, % des masses d'eau sont en bon état. On est obligé de fermer des captages, non pas parce qu'il n'y a plus d'eau. Mais parce qu'ils sont impropres à la consommation métal au chlore. Des plans nitrate. Algues vertes qui se succèdent d'année après année sans aucun résultat. Donc il y a un moment effectivement on peut dire que le marché que l'économie est au-dessus de la biosphère mais je crois qu'on se fait un peu rattrapé par la patrouille. Et je suis triste de voir que malgré toutes les alertes. On a bien vu pour le GIEC, les les les rapports se sont empilés sur la biodiversité et les rapports s'empilent également et on est toujours en train de foncer dans le mur parce qu'il y a le sacro-saint marché qui est au-dessus de tout et qui est la norme absolue et moi je pense que, effectivement, on est là dans une impasse et qu'il faut un jour un moment se poser les vraies questions. Merci, cher collègue, la parole est à madame Patricia Schillinger pour le groupe RDPI pour six minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Avec 70 milliards d'euros d'exportations en matière agricole et agroalimentaire. La France demeure un grand pays d'agriculture elle reste au niveau européen, le principal producteur loin devant l'Allemagne et l'Italie. Pourtant le rapport dont nous débattons ce soir dresse un constat alarmant. La ferme France serait en déclin. Si nous pouvons être en désaccord avec un certain nombre de préconisations de ce rapport. Je tiens néanmoins à en reconnaître et saluer la grande qualité de ce point de vue je remercie les rapporteurs pour leur travail. Ceci étant, le rapport pointe du doigt la montée en gamme promue par les pouvoirs publics, elle mettrait en péril en péril notre potentiel productif rendrait l'alimentation d'origine française inaccessible aux plus modestes sans pour autant favoriser son exportation tandis qu'au contraire on assisterait à une explosion d'importation. La France serait ainsi coupable, coupable d'avoir sacrifié la compétitivité de son agriculture au profit de sa montée en gamme coupable de privilégier la qualité de son alimentation à la quantité, que semble ainsi posé en filigramme ce rapport et celle dépassé selon moi du choix entre production de masse et productions de qualité, quand il nous faudrait plutôt nous interroger sur les moyens de concilier ces 2 objectifs le secteur agricole et aujourd'hui au Carrefour de ne nombreux enjeux dont il ne peut faire. Abstraction en plus de devoir certes assurer la souveraineté alimentaire de notre pays, il doit répondre à une exigence croissante de qualité et s'orienter vers des pratiques plus durables soucieuse du climat. Cela correspond à une attente sociétale forte qu'aussi bien le monde agricole que le politique ne peuvent ignorer, constitue constituent également la condition de la survie et de la pérennité même de la ferme France aussi dissocier combien nous produisons de comment nous produisons conduirait hein Macron immanquablement à revenir sur les nombreuses transition engagée et en plus de sa compétitivité mettrait en paix Evry le notre modèle agricole lui-même alors que les contraintes qu'une rencontrent nos agriculteurs sont déjà nombreuses rejoindre à ces Angers suppose il est vrai d'importants efforts de leur part qui à défaut d'accompagnement grèverait considérablement leur compétitivité. Car si l'on demande aux agriculteurs de s'adapter d'anticiper les bouleversements qu'engendre le changement climatique, c'est avant tout pour leur permettent de dépasser ces bouleversements la survie et la pérennité de notre modèle agricole sont donc au coeur de la politique du gouvernement et c'est notamment pour mieux protéger les agriculteurs face à des ces changements et leurs conséquences, qui a été réformé l'assurance récolte, ce sont ainsi près de 560 millions qui ont sont consacrés accompagner les agriculteurs le sont aussi dans le un cadre européen ce grain Khadr permet à nos agriculteurs non seulement d'emprunter la voie nécessaire des transitions mais de faire en préservant leur compéti il sécurise financièrement les agriculteurs qui s'engage sur cette voie. À titre d'exemple, on peut souligner le soutien apporté au développement du bio par la nouvelle PAC avec pas moins de 340 millions d'euros en moyenne par an. contribue plus largement à établir les bases d'une concurrence équitable entre les États membres. La France a ainsi profiter de sa présidence de l'Union européenne pour faire de la question de la réciprocité des normes un impératif. Le rapport dresse donc un bilan juste et sans appel des politiques menées depuis les années 90 mais occulte toutefois le tournant pris depuis 2017 pour renforcer notre agriculture soutenir nos agriculteurs, dans leur transition et préparer la ferme 2030 préparer la ferme France de demain passe par l'investissement c'est tout d'abord investir pour innover avec le plan France relance et France 2030, ce sont plus de 4 milliards d'euros investis C'est ensuite investir pour produire en quantité et en qualité ce sont ainsi 150 millions d'euros mobilisé pour le cadre du plan. C'est aussi la mise en oeuvre du plan de souveraineté pour la filière fruits et légumes pour qu'elle augmente sa production, préparer la ferme France de demain c'est sécuriser les revenus agricoles et garantir à nos agriculteurs des prix rémunérateurs depuis la loi Egalim hein. nous faisons de la question de revenus agricoles, une priorité. Préparer la ferme France de demain, c'est veiller à l'accès de tous, dont les ménages les plus modestes à une alimentation de qualité. Le chèque alimentation durable ou encore les dispositions adaptées dans la loi Egalim et dans la loi climat vont dans ce sens. Préparer la ferme France de demain s'éveiller au renouvellement des générations. Cela passe par la formation, le soutien à la transition et à l'installation, car il n'y a pas de ferme France sans agriculteurs face à ces nombreux chantiers l'État plus que jamais se doit d'accompagner de soutenir les acteurs dans la transformation, c'est le sens de l'action que mène la majorité au côté du gouvernement, donc lui au choc des. Compétitivité oui au soutien à l'export mais sans pour autant renier notre ambition pour une agriculture Agriculture plus innovante durables et performantes. Je vous remercie. avons essayé de mettre en oeuvre depuis 5 ans, 6 ans bientôt. D'abord reconnaître que le chemin est assez long hein, pour retrouver la souveraineté de la compétitivité parce que c'est. Et je sais plus qui, tout à l'heure disait, vous n'êtes pas forcément comptable je me considère comme au fond comptable de ce qu'on a fait depuis 30 ans parce que ce serait trop facile de dire c'est la faute des autres. Je pense qu'il faut qu'on essaie chacun de faire. Notre part du chemin. Vous avez je voudrais souligner simplement 3 points. D'abord la place importante qu'on doit donner à l'innovation, à la recherche. À l'expérimentation parce qu'on a besoin de trouver, y compris en termes de transition. Et de convaincre les agriculteurs que c'est par cette voie là qu'on essaiera de trouver des solutions, des alternatives par exemple aux produits phytosanitaires par exemple à la sortie d'un certain nombre de produits phytosanitaires parce que il y a que ce moyen là qui permettra de faire des choses qui nous permettent par ailleurs de garantir notre souveraineté notre compétitivité 2ème élément, vous avez été. Qu'est ce qu'on a fait ce qui a été votée d'ailleurs au Sénat avec grâce aux travaux. Vous avez mené ici au Sénat sur le système assurantiel. Je pense qu'on a un dispositif qui est un début positif solide. L'assurance est à la fois le dispositif assurantiel qu'on a qu'on a voté qu'on a produit. Mais c'est aussi d'autres facteurs, l'assurance, c'est la capacité qu'on a de donner aux agriculteurs, que le système sur lequel il s'installe. C'est un système qui dans 30 ans sera résiliée en résistant en particulier aux questions dérèglement climatique aux grandes transitions qui sont à l'heure, c'est-à-dire la question de l'accès à l'eau, c'est-à-dire la question de la modification des pratiques, c'est-à-dire parfois d'un certain nombre de systèmes qui vont évoluer parce que un degrés de température c'est le climat de monsieur le sénateur. De Toulouse à Rennes et le climat Toulouse à Rennes ça change la production à Rennes et ça change la production à Toulouse, donc si on ne le dit pas aux agriculteurs, y compris dans les installations ferait défaut à notre responsabilité, je crois que pour le coup, nous le partageons de transition qu'il faut faire question c'est la transition dans cette affaire-là et pas dire simplement, c'est facile, je, je, non j'ai pas dit que vous disiez ça, parce que je pense qu'il faut qu'on qu'on assume le fait qu'on a besoin réellement de transition et les transitions c'est du temps parce que c'est des facteurs de production et c'est aussi des facteurs humains qu'il faut accompagner dans cette affaire et puis 3ème élément. Vous avez évoqué la question européenne. Je pense qu'il y a un certain nombre de débats. Moi je suis pour qu'on mette ces débats-là, y compris les débats souveraineté parce que c'est un débat important à l'aune de ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine et le Covid au niveau européen parce que c'est là qu'on réglera les problèmes aussi. Si Monsieur le Ministre, la parole est à monsieur Serge Mérillat ou pour le groupe socialiste, écologiste républicains pour 9 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, madame la présidente de la commission je je voudrais en préambule, avoir une pensée pour notre collègue Jean-Claude Tissot qui est pour nous. Chef de file de l'agriculture qui est. Confronté à un drame personnel et donc. Au pied levé, j'ai repris, j'ai repris son intervention et donc. J'ai pris les 9 minutes qu'on ne devait se partager. J'allais dire en introduction de ce débat. Notre rapport a fait un constat sans appel qui vient d'être dit par beaucoup d'intervenants. La ferme France décline partout sur nos territoires. Les agriculteurs nous interpelle nous font part des difficultés parfois insurmontables. Pour celles et ceux qui nous nourrissent et ne sont pas rémunérés à hauteur de leur engagement. Notre agriculture, notre gastronomie sont réputés dans le monde entier la qualité de nos denrées notre savoir-faire ne sont plus à démontrer. Pourtant à l'heure où le commerce international de produits agroalimentaires n'a jamais été aussi dynamiques. Nous ne sommes pas au rendez-vous. Nous sommes le seul grand pays agricole dans les parts de marché recule quand dans le même temps nos importations de produits agricoles. en 20 ans, nous sommes passés de 2ème à 5ème exportateur mondial notre excédent commercial n'est essentiellement tirée que par l'effet prix de nos amis, nos, nos exportations notamment des vins et spiritueux. Filière d'ailleurs de plus en plus concurrencé. Mes chers collègues, cette situation doit nous inquiéter nous inquiète dans un contexte géopolitique tendu couplée à une inflation galopante, nous le constatons les prix des denrées alimentaires s'envolent et certaines viennent à manquer. Plus que jamais, nous devons repenser notre modèle agricole pour tendre vers la souveraineté alimentaire pour ne pas être dépendant de l'extérieur pour notre alimentation et il n'y a rien de pire que les peuples qui ont enfin. Nous devons pouvoir être en mesure de nourrir convenablement les Français quelle que soit leur classe sociale. Nous devons probablement reconnecter la l'agriculture avec des attentes des consommateurs. Notre pays, grande puissance agricole le grenier de l'Europe. Le peut, sous réserve d'une réelle volonté politique pour ce faire, il est impératif de réarmer la ferme France en lui donnant les moyens de ses ambitions en lui donnant les moyens d'être compétitive redevenir compétitif. C'est d'abord redevenir attractif aujourd'hui face aux difficultés financières, matérielles ou techniques, beaucoup d'agriculteurs ne s'en sortent plus. Précarité et agree bashing n'incite pas à l'installation de nouveaux exploitants en ce sens. Les chiffres publiés par la MSA ces dernières années sont éloquents et de voix et doivent nous inquiéter. Réforme de l'enseignement du foncier juste rémunération des agriculteurs ou encore revalorisation des retraites agricoles les chantiers sont nombreux et les embrasser à la matière ne sommes pas pour l'heure suffisante. Redevenir compétitif si signifie aussi revoir nos politiques agricoles passer. La stratégie insufflé par le président de la République lors du discours de Rungis et il y a pour objectif la seule montée en gamme. Ne peut pas être l'Alpha et l'oméga de notre agriculture d'autant plus que les agriculteurs en vu le montant de leurs charges s'envoler la fiscalité augmenter la concurrence mondiale, se développer et ont pu constater un soutien pour le moins mitigé du gouvernement dans les accords de libre-échange. Faute d'un accompagnement adapté et à la hauteur des ambitions du président de la République. Cette stratégie du tout montée en gamme risque d'entraîner notre pays dans une crise de souveraineté alimentaire et de pouvoir d'achat. Pour faire face à la demande et redonner une dynamique à notre ferme France nous devons j'en suis convaincu. Réinvestir le marché coeur de gamme et boosté notre productivité, l'agriculture française est capable de répondre à ces défis nos éleveurs, nos agriculteurs sont responsables et soucieux de produire des denrées de qualité faisant leur davantage confiance et surtout

C'est le grand défi des 10 années à venir hein. Jeu environnementaux, gestion de l'eau. Concurrence internationale déloyale par des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes, il est urgent de sous. Sauvegarder notre souveraineté alimentaire pour ne pas de mettre totalement dépendants des aléas géopolitiques sanitaire ou encore climatique les trois années que nous voulons traverser ont été dur mais ont été également riche un anciennement. À l'enseignement. Il est temps de reconquérir dans tous les domaines notre appareil productif et cesser de s'en remettre aveuglément aux sirènes de la mondialisation à tout va. Il n'a pas pour but d'opposer les modèles agricoles et les agriculteurs entre surtout pas, il n'a pas pour but d'opposer le conventionnel et le bio d'opposer les céréaliers et les éleveurs l'agriculture dite productive encore faut l'faudrait le définir et celle plus familiale etc Il faut produire pour toutes et tous dans un cadre clair afin de répondre aux atteintes diverses de nos concitoyens d'avoir une alimentation sûre de qualité local diversifiée mais également accessible économiquement. Ce dernier point été essentiel pour que chacun de nos concitoyens puissent manger français, tous les jours et pas uniquement lors du repas du dimanche. Rappelons-nous que le contenu de l'assiette et le 1er révélateur d'inégalités. Mes chers collègues. Pour ce faire nous devons changer de cap, mais non sans garde-fous. En tant que co-repart co-rapporteur socialiste d'un rapport transpartisan. J'ai fait part à mes collègues de divergences à l'égard de certaines propositions La la richesse de la confrontation d'idées si on est entre nous. On sera d'accord entre entre nous mais il n'en sortira pas grand-chose et et et c'est intéressant de se confronter de partager et et de trouver des accords pour avancer. les dans les divergences. Je pense notamment à l'évolution du rôle qui pourrait donner à la ne cesse. La rentabilité et la compétitivité de notre ferme France ne doivent pas altérer la qualité des produits, constituer un risque pour la santé de nos concitoyens, c'est bien évidemment la ligne rouge et il en va de même pour la réduction des coûts coûts de production qui ne peut pas prendre à la forme d'une détérioration des conditions salariales des travailleurs. Nous avons échangé et sur ce point là bien sûr, nous avons trouvé des accords. Monsieur le Ministre ce rapport transpartisan est une contribution qui me semble pertinence face à l'état de notre modèle agricole. L'accueil positif qui lui a été réservé par le monde agricole en témoigne.

mais il doit être accompagné par une présence de l'agriculture française dans tous les segments du marché et c'est ça, à mon sens l'enjeu. le groupe politique auquel j'appartiens a d'ailleurs été à l'origine de nombreuses initiatives lorsque nous étions en responsabilité, je pense notamment à l'engagement de Stéphane Le Foll, en matière de développement du bio et de l'agro-écologie ou encore celui des sénateurs de mon groupe depuis des années en faveur du développement des paiements pour services environnementaux. Ces modes de production, de distribution de mise en valeur des produits nord-terroir je les encourage dans mon département, nous devons collectivement les encourager. Je l'ai dit, la stratégie de montée en gamme nécessite un accompagnement fort et massif des agriculteurs pour limiter la différence de prix sur les étals. L'objectif doit être la démocratisation de ces produits, afin que chacun puisse en bénéficier. Mais pour l'heure, monsieur le ministre à la priorité de nourrir tous les Français et que tous les Français et les moyens de se nourrir. Et nous ne sommes pas sur le bon chemin, rendant à nos agriculteurs. La fierté de produire et n'oublions pas que dans nos départements ruraux. L'agriculture est souvent la dernière activité économique qui remplit sans contrepartie financière, un rôle irremplaçable dans l'aménagement et et l'entretien de l'espace. mais Riou. J'essaierai de répression dans mon propos conclusif. Mais vous avez dit d'abord, il y a rien de pire. Vous avez raison. Que que de ne pas être en capacité de pouvoir nourrir son propre propre peuple. C'est ce n'est pas principalement un sujet français mais c'est un sujet qu'on a à l'avenir en particulier lié au dérèglement climatique. Donc on doit veiller à cette question, vous avez tout à fait raison. De pouvoir être en capacité de continuer à pouvoir nourrir notre propre peuple parce que c'est une question de coût de souveraineté essentiel et on sait bien que les grandes crises. Sociales et grande crise révolutionnaire et il y a pas besoin de remonter en 1789. De l'autre côté de la Méditerranée un ont vu, elles viennent souvent de crise alimentaire. Donc c'est un sujet de stabilité. Pour nos pays et c'est un sujet de de stabilité pour les pays qui sont à nos frontières. Donc on a besoin de s'assurer de notre souveraineté et de la souveraineté des pays tiers parce que sinon c'est une déstabilisation globale et donc je partage cet élément-là 2ème élément. Vous avez évoqué la question et des attentes et des besoins des consommateurs. Oui on a besoin de travailler sur un certain nombre de nos concitoyens qui ne peuvent pas accéder à une alimentation parfois de qualité ou parfois une alimentation diversifiée. C'est la suite, c'est le travail que nous devons poursuivre. Sur la question du chèque alimentaire et du chèque alimentation parce qu'effectivement là on a un sujet. en partie dans le rapport. Elles sont diverses et donc il en a besoin d'une diversité des productions et d'une diversité de l'offre pour les consommateurs. De la moyenne gamme du haut de gamme et de la et et l'entrée de gamme et c'est à ça qu'il faut répondre parce que les consommateurs ils ont des besoins et des attentes diverses. Vous disiez la stratégie. Comme si la stratégie de montée en gamme sur sur les centaines et centaines de signes de qualité. Pensez qu'il y en a combien qui ont été créés ces 5 dernières années. Ça fait 70 ans qu'on des, enfin 60 ans qu'on développe de signes de qualité, enfin je veux dire c'est pas une nouveauté, les signes de qualité c'est pas le discours de Rungis était venu dire que c'était une capacité à portée de la rémunération. Assumons collectivement et c'est plutôt une fierté que les signes de qualité, nous les avons portée. Chez nous. Et à l'extérieur de nos frontières, parce que nous avons fait reconnaître y compris dans les accords internationaux et ils sont que dans la marque France que nous avons à défendre cette question de la qualité, elle est une question de la marque France et on a beaucoup exporté parce que nous avions. en partage une identité un Patrimoine une culture et de la qualité et donc il ne faut pas complètement s'en délester, vous l'avez pas dit d'ailleurs mais y compris en terme d'export. Oui, Monsieur le Ministre, la parole est à madame Françoise Ferrat pour le groupe Union centriste pour 4 minutes. Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission. Mes chers collègues. je ne vais pas répéter ici les conclusions de nos brillants rapporteur messieurs du plomb, l'eau et Riou. Mais il faut nous rendre à l'évidence, notre excédent commercial agricole s'érode et nous perdons en compétitivité. Le Sénat formule 24 recommandations afin d'y remédier à l'horizon 2028. Heureusement la France demeure une grande puissance agricole et garde de son rang de principal producteur européen. Devant l'Allemagne et l'Italie. Néanmoins, en 20 ans cela déjà été dit, la France est passée du 2ème rang ou 5ème rang mondial. Je pourrais me satisfaire de cette situation, il me dire que finalement on ne s'en sort pas si mal. Mais Monsieur le Ministre, ce serait nier plus de 20 ans de travail au Sénat et de rencontres avec les organisations agricoles. Ce serait nier le rapport parlementaire que j'ai menée avec Henri Cabanel sur le suicide des agriculteurs. Ce serait nier, monsieur le Ministre, 6 années de rapports budgétaires et d'auditions au cours desquelles nous faisions le constat d'une perte de compétitivité des exploitations françaises. Bien souvent du fait de surtransposition de normes européennes ou de contraintes que j'appelle administre Atos paf raciale et qui vont, qui plombe la vivacité de nos fermes. Pour illustrer mes inquiétudes et des alertes je rappelle qu'en 2021. Le solde commercial français s'élève à 8 milliards d'euros. Ces 3,4% de plus qu'en 2019. D'accord et principalement en raison des exportations des vins et spiritueux dont le solde s'élève à 14,2 milliards d'euros. Ce secteur constitue le fleuron d'un secteur agroalimentaire qui n'arrive pas à valoriser correctement le reste de ses produits. En clair, sans les vins nous serions déficitaires. Cela ne choque pas hein c'est un État surendetté mais permettez-moi de lettres. À qui et à quoi attribuer cette perte de compétitivité. Peut être la stratégie du tout monter en gamme menée par votre majorité depuis 2017. Nous rapporteurs citent le poulet du dimanche. Ainsi, les Français se tournent vers la découpe les produits élaborés, dont 16% seulement proviennent des Sico. Le marché important du poulet standard et donc ouvert aux importations et presque un poulet sur Dieu est importé, contre 20% en 2000. Je peux citer les betteraves qui se trouve coincés par la justice européenne. Mais rassurez-vous le Brésil sera nous ventre du sucre pour pas cher, à des conditions déplorables pour l'environnement et le droit social. Je citerai le coût de la main d'oeuvre qui est de une à 3 fois plus élevé qu'en Espagne, Allemagne ou Pologne. Je pourrais multiplier les exemples de surtransposition des normes européennes. En effet, notre pays se caractérise par la place importante des surtranspositions politique ou l'arbitrage politique l'emporte sur le choix d'une transposition mesurer. D'autres pays se sont également poser cette question. Il ressort que la majorité des États afficher une part de normes d'origine européenne plus faible que nous. 14% pour le Danemark 10% pour l'Autriche. Je vous accorde 39% pour l'Allemagne souhaite. Mais pour contrer ce poids l'Allemagne suit depuis 2015 l'impact pour ces entreprises de la législation européenne et a adopté le principe du One I One out pour contenir la complexité.

Il vous faut faire le bilan de 20 années de stratégie agricole pour quel résultat stoppons le déclassement international il est encore temps d'inverser la tendance. Écoutez, le Sénat, Monsieur le Ministre, ils les échos de la ruralité et de nos agriculteurs. Je vous remercie. Merci, cher collègue, Monsieur le Ministre.

Aussi quotidiennement possible ou hebdomadaires que possible. Plusieurs éléments, vous dites. Vous ne vous satisfaisaient pas. Pas de la réunion de l'arrêt de la situation. Moi non plus, en plus je suis passé satisfait de la situation en termes de souveraineté de la ferme France vous l'avez rappelé, c'est des dizaines d'années. Au fond on a laissé faire les choses sans regarder dans le détail, c'est petit à petit, que les choses sont faites, il y a pas de grande rupture en fait vous regardez c'est une tendance assez lourde. Oui non. Et donc on a besoin de retisser la même chose que ça ne sera pas une courbe à verser. On a besoin de faire avec patience avec modestie chacun notre Oeuvres. Dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent et les années qui viennent pour essayer de reconstruire patiemment la souveraineté que nous avons perdu 2ème élément, vous êtes dans un département, vous avez parlé d'un fleuron qui est la la viticulture. Alors d'abord je signale que ce n'est pas inintéressant de dire que. Effectivement c'est la viticulture. Alors vous dites c'est un fleuron. Je pense que la filière. Animale est un fleuron que la filière végétale pourrait être un fleuron et fond simplement la viticulture et ce qui reste d'émergeant des fleurons français mais nous avons plein de fleurons et en fait, nous avons besoin de renouer avec ça je signale juste que la viticulture et c'est le seul élément d'export qui soit totalement sous la belle des signes de qualité. Donc c'est pas complètement inintéressant dans la démarche export de penser que l'usine de qualité pour l'export en tout cas ça a une vocation intéressante et vous en savez quelque chose dans la mort. Et puis 3ème élément vous avez évoqué, vous avez raison, la question. De l'espace européen des des normes que nous nous infligeons nous-mêmes français quand d'autres ne s'impose pas les mêmes et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, je pense que nous avons besoin de réfléchir en européens et avec les autres collègues européens à la façon dont nous avons envie de normer d'évoluer sur un certain nombre de transition qui sont nécessaires et nous avons besoin de réfléchir au niveau français aussi sur ce qu'est la question des transpositions des surtransposition et parfois aussi de la sur administration qui n'est pas une forme c'est pas de la surtransposition ça c'est la façon dont on gère. Des politiques publiques. Reconnaissons que ça je me méfie toujours des ministres-qui disent on va essayer de simplifier parce que généralement c'est au bout de la du tube, c'est plus compliqué. Donc il faut le faire aussi avec modestie mais vous trouverez sur ce chemin-là et merci du travail que vous faites aussi pour essayer de regarder, là on peut pratiquement essayer de simplifier les choses. Merci, monsieur le Ministre, la parole est à madame Béatrice Gosselin pour le groupe Les Républicains pour cinq minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Au mois de septembre 2022, le journal Le Point écrivez. La commission des affaires économiques du Sénat tirent pour la nième fois le signal d'alarme. La ferme France ne va pas bien, elle produit de moins en moins et pour nourrir le peuple France des importations explosent. Notre pays aux Terres fertiles au climat tempéré au savoir-faire et à la diversité des produits à de nombreux atouts pour réussir. Pourtant notre agriculture va mal et le monde agricole est préoccupé par un certain nombre de points au nombre desquels figurent des changements réglementaires permanent ainsi que la pression concurrentielle croissante, la compétitivité de notre agriculture chutent et les conséquences sont inquiétantes pour l'instant sous souveraineté alimentaire. Beaucoup de filières souffrent et certains certains succès cache bien des problèmes. 2ème, producteur de lait de l'Europe, la France alimente son marché intérieur avec 60 58 % de sa collecte tout en exportant 40% de sa production en majorité vers les pays européens. En Normandie, la filière lait détient un troupeau de 547.000 vaches laitières en 2021. Pourtant si les éleveurs maintiennent les produits laitiers. Sur la scène internationale c'est au prix de la faiblesse de leurs revenus pour répondre à la guerre des prix. Ce soi-disant miracle français se traduit plutôt par filière en danger et désastre annoncé pour la production laitière en effet le manque de trésorerie pénalise les investissements susceptibles d'améliorer la la productivité et les revenus. Des exploitants agricoles découragés par les revenus faibles. Le coût des investissements et les contraintes quotidiennes de l'élevage arrête la production laitière ainsi pour la Normandie c'est une baisse de 32% de 2010 à 2020 et des régions de bocages et d'élevage comme la Manche voient leur cheptel bovin diminuer de façon importante. C'est une situation de plus en plus difficile à supporter pour les producteurs et un point de blocage pour les jeunes candidats à l'installation. Se pose alors le problème de la transmission. Sachant qu'un éleveur sur 2 à 50 ans ou plus et que la baisse du nombre d'exploitations laitières et la plus importante en France que dans les autres pays européens. Le nombre d'élevages de porcs a chuté de 40% en 10 ans en Normandie. La filière porcine est une production exigeante sur le plan technique est très aléatoire sur le plan économique, le prix de ventre fuck fluctuent énormément alors que les charges continuent de progresser. La production porcine française et donc plutôt à la baisse et dans le même temps en Espagne 1er producteur européen 58 millions de porcs ont été abattus en 2021. Dans un autre domaine, la production française de pommes a été divisé par 2 depuis 30 ans on en exporte devant moins qu'il y a 7 ans alors qu'une pomme sur 3 est importé pour être transformé. La surtransposition des normes nuit également à l'agriculture française pour qu'elle soit plus compétitive. La France importe impose des normes plus contraignantes que les directives européennes, ce qui augmente le coût de production par exemple la France oblige à recyclage des eaux issues de la transformation laitière alors que les pays concurrents sont autorisés à réutiliser ces eaux sans traitement. L'État français interdit 145 produits phytosanitaires pourtant utilisé en agriculture dans les pays concurrents, concurrent de l'Union européenne. Cela crée cette distorsion de concurrence évidente. Les produits issus de l'agriculture française sont souvent plus chers pour les consommateurs, notamment en raison de l'importance des charges dont le coût de la main-d'oeuvre qui est le plus élevé en France qui est plus élevé en France. Pardon. Depuis 2017, dès son discours de Rungis. Le président Macron prône le tout monter en gamme et même si cette stratégie répond à certains marchés cela n'améliore pas globalement la situation. Pour les exportateurs et consommateurs nationaux le positionnement français haut de gamme ne justifie pas un tel écart de prix avec les concurrents les habitudes de consommation des ménages se traduisent en fait par une réduction des quantités achetées au regard des prix. La pomme bio par exemple qui revient en moyenne à 2 fois plus cher que la pomme conditionnel est acheté par seulement 21% des consommateurs. Elle est également difficile à écouler à l'étranger donc 38% des producteurs bio sont donc obligés à écouler leur surproduction sur le marché conventionnel, soit une baisse de de de revenu de 820 euros par tonne. Nous devons désormais agir avec force pour éviter que notre pays à la terre nourricière devienne un pays sans autonomie anime alimentaire le rapport sénatorial a formulé plusieurs recommandations en ce sens pour maîtriser notamment des charges de production, éviter les surtranspositions et relancer la croissance de la et de la productivité je installé le qualité du travail réalisé et souscrit pleinement ses recommandations. Nous devons absolument engager au plus vite ce choc de compétitivité, notre pays manque de stratégie. Or la clé de la réussite des pays qui gagne, c'est leur capacité à devenir à définir une stratégie et un objectif clair la compétitivité doit être un objectif politique clair. Nous le devons à notre agriculture dans cette activité est au coeur de l'avenir de nos territoires que le Sénat a précisément vocation à représenter, je vous remercie. Merci monsieur le président. Merci madame la sénatrice Gosselin. Vous avez évoqué un certain nombre de filières. Vous avez d'abord évoqué c'est normal compte tenu de votre région les. Les filières d'élevage.

Et on devrait regarder les modèles d'élevage qu'on a construit en France que c'est un modèle qui à bien des égards et quand j'entends un certain nombre de gens nous parler d'agro. Non mais c'est c'est pour aller dans votre sens, de gens qui nous parle. D'agro-industrie d'élevage industriel des fermes usines. Enfin faut qu'ils aillent à l'extérieur de nos frontières et il y a pas besoin d'aller en Chine. Faut aller parfois très près pour voir la vers la réalité des élevages et donc on ne devrait plutôt se féliciter d'avoir le modèle d'élevage que nous avons. Parce que ça c'est un facteur y compris d'attractivité pour les meetings. 2ème élément sur l'élevage, je fais un petit zoom sur le lait, vous avez raison, on a un sujet particulier sur le lait et la question de la rémunération et la question des conditions de travail. La question du portage des capitaux parce que c'est des capitaux qui sont forcément assez lourd pour un jeune, y compris dans un modèle de dérèglement. Et globalement sur l'élevage, on a pensé à vous pensez le système. Différent pour les Normands pour les Bretons est différent pour les Bretons que pour les éleveurs du Massif Central, cher à Monsieur ce n'est pas le même modèle parce que ça n'est pas les mêmes qu'on s'constante pédo-climatiques ne ce ne sera pas le même élevage. Et donc il faut qu'on essaie de travailler, ça. Donc c'est un élément qui est un peu vous avez évoqué la question quel est le le le comment on essaie de de dire ce qu'on veut faire, à mon avis, c'est la question de la souveraineté au coeur de notre de notre fini grade. C'est ce qu'on va essayer de faire et de développer et je viendrai bien volontiers, vous vous en parler sur le plan de souveraineté, fruits et légumes c'est de travailler sur la question des phytosanitaires la réduction et les alternatives c'est la question des investissements dont on a besoin pour faire face aux défis demain, c'est la question de la main d'oeuvre et comment on gère cette question là. Pour retrouver de la compétitivité. C'est la question de retrouver des filières d'excellence et de répondre aux besoins des consommateurs. C'est comme ça qu'on essaiera et qu'on réussira à faire un certain nombre de choses, on doit aller. Il me semble que c'est comme ça qu'on arrivera à faire, secteur par secteur et j'allais dire presque filière par filière. Merci, monsieur le Ministre, la parole à monsieur Christian Klinger pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En lisant ce rapport, je me suis souvenu des leçons que j'apprenais plus jeune. La France était alors le grenier à blé de l'Europe un pays de cocagne. 2ème exportateur mondial. Aujourd'hui nous sommes cinquièmes dans les années 80 il y avait 1,2 millions d'exploitations agricoles, aujourd'hui on en compte un peu moins de 440.000. Oui, en 2023, la France est l'un des seuls grands pays agricoles, dont les parts de marché recule, tandis que ses importations alimentaires explosent le potentiel productif agricole s'érode d'année en année. Baisse du nombre d'exploitations, chute de la surface agricole utile en culture et plafonnement des rendements la productivité de l'agroalimentaire, faute d'investissements suffisants est également en berne. Nos collègues ont donc passé plusieurs mois à dresser un tableau exhaustif de la filière agricole mais plus intéressant. Ils se sont penchés sur les causes et donc ont interrogé l'esprit des réformes successives qui ont conduit notre agriculture aller aussi mal. Depuis plusieurs décennies, nous nous sommes habitués à entendre une petite musique qui vitupère notre modèle agricole. Pourtant l'un des plus vertueux. C'est donc dans ce contexte politico-médiatique qu'en 2017 notre, notre président a plaidé pour la montée en gamme pour la montée en qualité la montée du bio. Les produits français n'étant plus compétitifs. Il fallait qu'il monte en gamme pour atteindre des marchés de niche qui serait plus rémunérateur et en même temps il allait ouvrir le marché aux produits étrangers. Coeur de gamme. Cette politique agricole à 2 faces sera une impasse. pot de lait et son pot au lait, ces décideurs ont rêvé. Adieu lait pommes tomates poulet oui comme Perrette ses gouvernements successifs ont fini par trébucher sur la réalité ce modèle était déconnectés des attentes des Français et des contraintes qui pèsent sur lui sont autant de boulets qui l'ont entravé. Ça se, c'est que, c'est ce que ce rapport très pédagogique démontre à travers notamment d'exemples tirés de la consommation quotidienne de nos concitoyens. Prenons l'exemple de la pomme. Il y a 10 ans. Nous en exportons 700.000 tonnes et importé ont 100.000 aujourd'hui. Nous n'en exportons plus que 350.000 et en importons 200.000. Derrière ces chiffres, ce sont nos pomiculteurs qui se sont adaptés à des contraintes toujours plus coûteuses pour produire la pomme parfaite mais pour la produire, on augmente son coût et les vilaines pomme manque. Pour les produits de transformation, comme le joue la compote. Les conséquences sont sans appel, la pomme française coûte un euros 18 à produire quand la pomme polonaise coup de 53 centimes. La consommation régulière de la pomme pourrait donc rapidement devenir un produit réservé aux consommateurs les plus aisés, laissant les pommes étrangères bourrés de substances interdites en France aux consommateurs les moins aisés et aux producteurs de produits transformés à base de pommes. Cette politique du tout monter en gamme a fait donc naître de risques majeurs. Une déconnexion totale de notre agriculture avec les attentes de nos concitoyens, lesquels connaissent une inflation alimentaire sans précédent et une crise de souveraineté alimentaire. La guerre russo-ukrainienne nous a rappelé l'importance géostratégique de larmes agricole. Certes, le ministère de l'Agriculture a été renommé corriger réellement le Tir est maintenant une nécessité. La stratégie farm to Forks qui nous entraîne vers la décroissance va à rebours de nos besoins et aujourd'hui se heurte à la situation géopolitique. À l'heure où nous découvrons le prix de la dépendance énergétique. Comment pouvons-nous, ne pas doter la France d'une agriculture souveraine et compétitive. Nous ne pouvons plus nous acheter une bonne conscience environnementale sur le dos de nos agriculteurs. Ce serait irresponsable vis-à-vis de nos enfants. Ce rapport ne donne les clés pour redresser la barre de notre filière agricole. Ce serait dommage de passer à côté. Merci et ne de pas les mettre en oeuvre. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Sénateur merci. Vous avez évoqué plusieurs sujets. D'accord pour dire. Pardon, le discours du président de la République n'était pas dire tout monter en gamme. Mais simplement de dire que la montée en gamme et puis aussi un objectif et une perspective si on ne, de ne pas caricaturer et globalement la tendance collective que nous avons eu depuis 30 ans. C'est plutôt une volonté de monter en gamme. Donc faut qu'on essaye de le regarder comme ça, deuxièmement vous avez soulevé un point. Qui a été un peu soulevé ce soir mais je pense qu'il est un point important, c'est la question de la compétitivité de nos filières agro-alimentaire. On a des faux pas qu'on a un défaut de rémunération, on a un défaut de modernisation, on est en train d'y travailler, que le ministère de l'Économie et des Finances avec mon collègue Lescure de l'industrie parce qu'on a un sujet d'investissements dans les industries agroalimentaires qui est un sujet important parce que c'est un retard, y compris en retard en termes de compétitivité sur, sur lequel on, qu'on travaille, 3ème, élément de réponse, vous avez raison. La crise en Ukraine et vient de montrer que le le. L'alimentation c'est une arme. Et donc faut pas être naïf sur ces sujets-là et vous avez tout à fait raison, la souveraineté, c'est une question alimentaire, c'est une question de souveraineté tout court. C'est peut être la première des souverainetés que celle de pouvoir. Alimenter ça a été dit par le sénateur mairie ou je crois tout à l'heure que de pouvoir nourrir sa population et donc on a besoin de de le poser comme ça, y compris dans le débat public. C'est rien ne vaut mieux que de pouvoir nourrir sa population en termes de souveraineté et donc c'est comme ça qu'on pourra aussi avancer sur ce sujet. En revanche, juste un mot de dire. Je ne suis pas sûr que la question de la souveraineté soit complètement déliée du du défi environnemental le défi climatique. Le défilé grandes transitions. C'est aussi un défi de souveraineté parce que le modèle agricole. Il a ceci de particulier que lui il est dépendant du climat. Et que le sujet qu'on a sous les yeux, c'est un sujet de dérèglement climatique et donc ce n'est pas capable de, d'adapter notre modèle agricole au dérèglement climatique. Si on n'est pas capable de lutter contre le dérèglement climatique. À ce moment-là, c'est le modèle agricole lui-même qui sera en cause et c'est la souveraineté alimentaire qui sont en cause, donc c'est les deux, qu'on doit essayer de combiner, me semble-t-il parce que sinon il y a des modèles qui seront dans un, d'un, du fait du dérèglement climatique.

Merci monsieur le président, Mesdames, et messieurs les sénateurs, madame la présidente de la commission. D'abord vous dire le l'agent qui était la mienne au fond de pouvoir débattre, une nouvelle fois le sujet de la souveraineté alimentaire qui est un, un sujet qui est largement devant nous. Celui de la reconquête de cette souveraineté. Je voudrais vous êtes d'abord saluer le travail et la qualité du travail qui a fait le Sénat en particulier sur ce rapport mais globalement sur les sujets agricoles. Je ne dis pas par flagornerie, parce que je pense que souvent vous avez pu poser les débats avec le recul nécessaire sur des sujets qui sont des sujets beaucoup plus complexe que parfois la caricature. On est faite sur un certain nombre de tribune et dont je voudrais saluer le travail qui a été fait. Par le sénateur du plomb par le sénateur loué par le sénateur. Ce rapport sur la compétitivité. Le débat que nous avons eu ce soir sont utiles, me semble-t-il utile pour penser l'avenir de notre agriculture. Dans une période de défi. Ça a été dit par plusieurs d'entre vous et dans une période marquée effectivement par le conflit en Ukraine, qui demande s'il fallait encore en tout cas vous étiez-vous convaincu et moi aussi combien produire et nourrir. Produire pour nourrir ce sont des éléments essentiels. Ce rapport dresse des constats éclairant sur les politiques menées depuis la fin des années 90, notamment lorsque ses auteurs évoquent le choix de la stratégie de montée en gamme, cela montre que la perte de compétitivité à la caisse. Ce rapport conclut n'est pas un sujet nouveau j'évoquerai naturellement dans vos propos. Les orientations politiques que nous privilégions depuis 2017. Deuxièmement je voudrais partager avec vous que je voudrais partager avec vous, nous pouvons tout à fait, nous retrouver sur certains des constats formulés par le Sénat, y compris un certain nombre de solutions. Oui nous avons perdu des parts de marché à l'international. Sur certaines productions et la tâche est immense pour assurer notre souveraineté alimentaire. Pour autant, je ne crois pas qu'il faille opposer production de masse, je l'ai déjà dit et monter en gamme comme le fait ce rapport en considérant que la priorité doit aller à l'un. À l'endroit de l'autre. Si les deux qu'il faut faire pour répondent d'abord à la nécessité de répondre à la demande et aux besoins divers des consommateurs. Notre mission ne peut être de tout produire sur notre sol non plus ce n'est d'ailleurs pas le sens de la souveraineté alimentaire qui reposait sur un équilibre entre les productions, reconnaissons-le, des différentes régions du monde, ce ne serait pas réaliste, sachant que l'alimentation est aujourd'hui une affaire de complémentarité de compensation d'échanges saisonnier et aussi et encore plus sous forme de sous le régime des dérèglements climatiques. Tout l'enjeu est en réalité de combiner production de masse et monter en gamme selon des spécificités de certaines filières. Il s'agit d'un impératif pour maintenir la diversité de notre système de nos systèmes de l'école qui sont une forme et force c'est une richesse de combiner aussi la question de la souveraineté de la capacité à produire de la capacité à répondre aux besoins des consommateurs et aussi de combiner les nécessaires transitions non pas seulement pour les transitions et ce qu'elle ce qu'elles sont une attendent parfois d'un certain nombre de nos concitoyens beaucoup nos concitoyens et parce qu'sont nécessaires à l'agriculture. Si on n'est pas capable d'adapter l'agriculture au défi du dérèglement climatique au défi parfois de la perte de biodiversité au défi du stockage du carbone dans le sol. On ferait défaut à la question de la souveraineté. La vérité c'est celle-là, il est à cet égard indispensable que nous accélérions la transition parce qu'du niveau d'exigence sera tout aussi essentiel pour la conquête de nouveaux marchés et la réponse à de nouvelles attentes. La question, c'est la question de la distorsion de concurrence qu'on peut se crée avec les autres États européens. Je voudrais conclure en indiquant ce qui a été fait depuis 2017. La question du revenu je y reviendrai pas autour des lois Egalim 1 1, égal M2 auquel vous avez largement participé. Vous aurez un nouveau texte. À établir mais je pense que nous avons, nous sommes mis sur le chemin. Demain, dit la présidente en commission si j'ai bien compris, nous sommes mis sur le chemin d'une inversion de la logique de la construction du prix, on n'est pas au bout de ce chemin-là. Mais pour la première fois on a posé depuis ce qui n'avait pas été posée depuis très longtemps, la question de la construction du prix elle doit démarrer des coûts de production. Deuxièmement, accompagner les transitions. Je l'ai dit au travers d'une Varenne agricole maintenant il faut le développer sur le territoire et le concrétiser sur le territoire. La question de l'accès à l'eau. Évidemment les adaptation au changement climatique. On essaie de porter au travers de France 2030 nous faisons enfin en sorte de défendre notre agriculture comme je l'ai dit tout au long de cette soirée en européen depuis la présidence française de l'Union. Oui nous avons inclus pour la première fois, l'idée, elle n'était pas du tout dans le débat public de réciprocité les clauses miroirs à l'intérieur des accords internationaux. Est-ce que c'est suffisamment fait aujourd'hui la réponse est non, mais c'est un travail quotidien que nous devons mener avec vous, avec les parlementaires avec les autres États membres de, de faire en sorte que ces clauses miroirs puisse s'appliquer et donc c'est sur ce chemin là qu'il faut se mettre pour faire en sorte que entre Européens, mais surtout avec. Les autres pays avec lesquels nous faisons du commerce un certain nombre de ces clauses puissent être défendu et respecté. Enfin, dernier point, je le dis en conclusion, vous dire que tout ça. Viendra aussi alimenter les débats que nous aurons au moment de la, du projet de loi. D'orientation et d'avenir de l'agriculture que j'aurai l'honneur de présenter. Dans les prochains mois, on est dans la phase de concertation elle vient poser l'ensemble de ces sujets. Le sujet de la rémunération. Le sujet des transitions le sujet des adaptations. Le sujet du portage du foncier. Le sujet du portage des capitaux. Le sujet de la formation et de l'innovation, c'est tous ces sujets-là qui feront, me semble-t-il. Pardon de l'expression. sûrement une forme d'éco-systèmes qui permettent finalement, on a beaucoup dit l'agriculture va mal et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de secteurs qui vont mal mais c'est un, un formidable métier qui porte du sens. Il y a beaucoup de voix à l'avenir parce que c'était une capacité à produire à nourrir à stocker du carbone à défendre un certain nombre de valeurs qui sont celles de notre territoire et donc c'est aussi ça qu'on essaiera au travers de cette loi. Merci à toutes et à tous de ce débat. Monsieur Laurent Duplomb. Au nom de la commission des affaires économiques pour cinq minutes. Et pour conclure ce débat. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre, ce n'est pas parce qu'on réécrit l'histoire qu'on en fait une vérité. La réalité c'est qu'en 2017 nous avions à la barre de la ferme France. Un président de la République qui disait pas tout à fait la même chose de ce qu'il dit aujourd'hui, comme d'ailleurs sur plein de sujets. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, le président de la République n'avait. Fait dans son discours de Rungis. Une déclaration qui était. Très claire et que le malheureusement beaucoup d'agriculteurs ou de représentants professionnels. N'ont pas su comprendre. Quand il parlait de la montée en gamme ce cher président de la République, Monsieur le Ministre. Il. En même temps. Le principe de dire. Que parce que nous n'étions plus compétitifs. Il fallait accepter que des produits viennent de l'extérieur. Tout temps. En organisant et en recentrant la totalité de nos véhicules notre agriculture sur la montée en gamme. Nous ne critiquons pas monsieur le ministre à travers notre rapport est bien que mes 2 autres collègues que je remercie. Nous ne critiquons pas la montée en gamme, nous ne critiquons pas les produits de qualité. Ce que nous critiquons. C'est la valse à 2 temps. C'est-à-dire le principe de dire d'un côté il faut que cette montée en gamme nous permettent de conserver une part d'agriculture, tout en acceptant politiquement. De laisser tomber des pans entiers de notre production. Et de l'autre côté de se gargariser à travers des messages tout fait d'agroécologie ainsi de suite. C'est ça la réalité du discours du président de la République de 2017 et je ne parle pas du discours de la Sorbonne. Monsieur le Ministre du même président de la République en 2018 qui était capable presque de vendre sur l'autel du sacrifice européen, la politique agricole pour la première fois. Dans l'histoire de France de la Vème République d'un président de la République d'abandonner la politique agricole pour c'est ça la réalité. Reprenez les discours et je demande à tous ceux qui ne les ont pas repris, reprenez le discours de Rungis, reprenez le discours de la Sorbonne. Tout ce que je viens de dire il y a dedans. Alors Monsieur le Ministre, la réalité c'est que la France décline. Elle décline et que la réalité de ce déclin, il s'explique par 70% liées à la productivité. Quatre grandes causes nous entraîne à cette baisse de près de productivité des charges plus élevées. Une main d'oeuvre à 5 fois plus cher qu'en Espagne, 1,7 fois plus cher qu'en Allemagne, 12 fois plus cher qu'en Pologne et une concurrence par exemple avec le Maroc et des heurts payés à 70 centimes. C'est une sur-transposition des normes mes collègues l'ont dit sans arrêt nous avons sans arrêt des normes françaises qui viennent encore améliorer amplifier le phénomène de normes de réglementation que les agriculteurs européens connaissent et que les Français sur augmente. La réalité de ces quatre causes, c'est aussi une guerre des prix certes que vous avez essayer d'endiguer par les différentes lois que vous avez mis en place mais qui consiste à faire qu'une chose, c'est qu'au bout du bout, nos industries agroalimentaires ne permettent pas de retirer suffisamment de bénéfices pour pouvoir réinvestir et est resté dans la course de la compétitivité, le 3ème cause de cette manque de productivité. C'est un état pas suffisamment protecteur. Monsieur le Ministre, combien d'exemples et en particulier la tomate. Nous avons laissé entraîner à à ce que ces productions qui sont faites dans d'autres pays puisse remplacer les nôtres la tomate marocaine qui au départ devait être de la tomate ronde finit par de la tomate grappe est amplifiée par la tomate cerise. Ce qui fait qu'au bout du bout, les seuls Français qui produisent des tomates sont quasiment condamnés à ne produire que des tomates anciennes. C'est ça la politique agricole qu'on veut demain. Le 4ème élément c'est climat médiatico-politique mes collègues l'ont dit, mais qui est catastrophique. Il n'y a pas un pays. Serge Merriot a donné l'exemple de l'Italie quand on va en Italie, on a l'impression d'avoir 58 millions d'ambassadeurs de l'agriculture italienne. Quand on est en France, on a 30 millions sur 67 de procureurs contre l'agriculture française. C'est ça, la réalité est que quand on a amplifié ces 3 phénomènes hé bien on se rend compte de quoi. On a 3. Conséquences, la première conséquence c'est qu'on perd notre souveraineté et pourtant tous les exemples sont en train de nous le donner et c'est pour ça que le président de la République a changé de ton et a changé de termes parce qu'entre 2017 à la mondialisation heureuse de multiculturalisme et tout ce qui était vendu comme étant le paradis sur terre par le Covid et par la problématique de l'Ukraine devient la souveraineté comme par hasard on redécouvre toutes les avantages de la souveraineté d'un pays qui est capable de produire et d'pays qui est capable de nourrir sa population le 2ème la 2ème. Conséquence de tout ça, c'est de diviser les Français en de la problématique de la montée en gamme, Monsieur le ministre, elle se caractérise par ça. La conséquence, c'est que vous avez un une partie relativement faible de la population qui peut avoir les moyens de se payer par, à travers son achat une agriculture qu'elle veut. Mais vous avez de l'autre côté et c'est ce que vous condamnez à faire tous les jours, la plupart des Français qui se retrouvent condamnés à n'utiliser et à ne n'acheter que des produits importés qui ne correspondent pas pour un tiers à nos normes ça veut dire en clair que nous sommes dans un jeu. Nous sommes dans un jeu qui a amplifié les phénomènes et qui fait qu'au bout du bout, la seule réalité c'est que nous interdisons chez nous et nous mettons dans le corner des productions pour finir par les manger par la porte de l'importation, c'est cela la réalité et les accords de libre-, échange, monsieur le président, si vous me permettez quelques secondes de plus. Les accords de libre-échange ne vont pas les changer. Est ce que vous savez aujourd'hui que la Commission européenne est en train de dire de de faire de partis sur les échanges. Les accords de libre-échange globaux qui seront soumis au vote des États membres et puis des accords de libre- échange.

Vous avez dépassé très largement, même plus que quelques secondes. Donc moi je mets un terme à votre intervention. Bon ben écoute je suis désolé mais mais il faut tenir dans les temps, c'est aussi quelque chose qui fait partie du règlement. Merci monsieur le président. Merci à vous monsieur le ministre et j'espère que vous comprendrez enfin qu'il faut faire quelque chose de bien pour notre et culture ne pas que le dire mais le faire. Merci, merci, cher collègue. Mes chers collègues, je vais lever la séance. La prochaine séance ce mercredi 8 février à 15h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.